La séance est ouverte.

j'ai reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 17 juin 2019 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 1 juillet 2019. Le décret vous a été communiqué.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une école de la confiance est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Monsieur le président, mes chers collègues, c'est une oeuvre de longue haleine qui va s'achever aujourd'hui par notre débat et, je l'espère, par l'adoption de ces nouvelles dispositions du règlement du Sénat. C'est une oeuvre de longue haleine dont l'ambition méticuleuse est de rendre notre règlement plus lisible, plus maniable, d'éliminer les scories, de regrouper dans les mêmes articles les dispositions qui s'attachent au règlement des mêmes problèmes,

entreprise de longue haleine a été conduite sous l'impulsion du président du Sénat, qui a naturellement veillé à la fois à la qualité et à la bonne organisation de nos travaux, mais aussi à ce que toutes les concertations nécessaires aient lieu avant qu'il ne dépose cette proposition de résolution. Nous engageons ce débat selon des modalités qui sont nouvelles, puisque c'est la première fois que la discussion sur l'évolution du règlement du Sénat se fait en partie selon la procédure nouvelle de la législation en commission.

Les réformes du règlement du Sénat ont toujours été inspirées par notre tradition de pluralisme sénatorial. Aussi sont-elles presque toujours assez consensuelles. J'ai pu vérifier, en auditionnant tous les présidents de groupe et tous les présidents de commission, que c'était une fois de plus le cas pour cette proposition de résolution. Je m'en réjouis, car nous sommes tous témoins des difficultés que, dans d'autres assemblées, la modification du règlement peut susciter entre les différents groupes. Nous sommes, il est vrai, beaucoup plus avancés que l'Assemblée nationale dans la modernisation de nos procédures. Je me réjouis de constater que beaucoup de dispositions adoptées au cours des années récentes, notamment ce qu'il est convenu d'appeler la « réforme Larcher » de 2015, ont constitué une source d'inspiration pour celle-ci : législation en commission, contrôle du respect du domaine de la loi et du règlement, droit de réplique pendant les questions d'actualité au Gouvernement. Le Sénat peut être fier de ses initiatives qui ont permis d'améliorer nos procédures, tout en respectant les droits des groupes minoritaires et d'opposition, initiatives qui aujourd'hui semblent devoir faire école. Malgré son volume, le texte que j'ai l'honneur de rapporter présente une portée volontairement limitée et un objectif beaucoup plus humble que les réformes de fond de notre règlement auxquelles nous avons déjà procédé ensemble. Cet objectif a beau être plus modeste, il est tout autant essentiel : il s'agit de clarifier, de simplifier et de codifier, bref de réécrire à droit quasi constant notre droit parlementaire pour le rendre enfin plus lisible. J'apprécie tout particulièrement de voir disparaître des dispositions du règlement que j'ignorais et qu'il a fallu exhumer pour l'occasion, car elles étaient tombées en désuétude. En cas d'urgence, par exemple, le règlement actuel prévoit que les délégations de vote sont faites par télégramme », avec l'obligation de transmettre une lettre de confirmation dans les cinq jours. Visiblement, les auteurs de notre règlement ignoraient tout des nouvelles technologies en usage au Sénat Notre règlement dispose également que les pétitions sont réunies au sein d'un « feuilleton », qui n'est plus publié depuis de très nombreuses années. Il mentionne encore des questions orales avec débat, mais celles-ci n'ont plus d'utilité depuis la création des débats d'initiative sénatoriale en 2009. Enfin, pour les scrutins publics, le règlement actuel prévoit que les secrétaires doivent se réunir- très précisément -dans le couloir droit de l'hémicycle pour les votes « pour » et dans le couloir gauche pour les votes « contre ce qui n'est pourtant plus le cas en pratique depuis longtemps. Cette disposition n'a donc pas de raison de subsister- n'est-ce pas, madame la présidente Assassi ? Certaines procédures sont également inutilement complexes, vous en conviendrez. C'est le cas, notamment, des mécanismes de « double annonce », monsieur Sueur,

Enfin, il y a parfois dans nos règles une forme de laconisme, de concision, qui peut paraître excessive et déboucher sur une certaine obscurité de nos procédures, procédures, lesquelles ne sont fixées qu'au travers de règles coutumières. Loin de vouloir absolument tout figer par des normes écrites, les plus importants de ces usages gagneraient à figurer expressément

tenir. Mon travail était déjà largement engagé par les travaux qui l'ont précédé. Je n'ai eu qu'à vérifier que la proposition de résolution se faisait bien à droit constant : j'en atteste. J'ai aussi été très soucieux de respecter l'esprit de cette modification du règlement. Nous pouvons, bien sûr, réfléchir à des évolutions plus profondes, même si celles auxquelles nous avons procédé sont encore très récentes puisqu'elles datent de 2015. en soit, si une réforme institutionnelle devait aboutir, il faudrait bien que nous en tirions les conséquences sur notre règlement. Le moment venu, nous aurons à nous poser tout un ensemble de questions. C'est la raison pour laquelle j'ai été très attentif à ne pas changer les équilibres profonds profonds et consensuels qui existent dans nos procédures parlementaires. J'ai néanmoins proposé quelques apports avec beaucoup de prudence et de précaution. La commission a bien voulu me suivre.

également que la commission ait consacré et précisé le rôle des présidents des commissions des finances et des affaires sociales dans le contrôle de recevabilité financière ou sociale, Nous avons aussi intégré la jurisprudence du Conseil constitutionnel- c'est déjà du droit positif, mais ça n'était pas du droit écrit -en ce qui concerne la tenue de jours supplémentaires de séance sur demande du Gouvernement. ailleurs, nous avons procédé à des clarifications techniques de procédure parlementaire concernant le vote par division et la seconde délibération. Nous avons adapté notre règlement à la mise en place du scrutin public électronique, prévue à compter du 1 octobre 2019, et pérennisé la mission de veille contre les « surtranspositions » confiée jusqu'à présent à la commission des affaires européennes à titre expérimental et qui n'a plus à démontrer sa pertinence. Je tiens, pour conclure, à saluer cet effort utile de clarification de nos règles. Il ne s'agit peut-être que d'une première étape, mais c'est une étape nécessaire. Il était judicieux de ne pas mélanger les genres et de s'appliquer à cet objectif de lisibilité, de maniabilité, de clarté, de modernité de notre règlement, avant d'entreprendre, le cas échéant, une révision plus

groupes. La parole est à M. Bernard Buis. Monsieur le président, mes chers collègues, nous sommes appelés à débattre d'une proposition de résolution visant à clarifier, à simplifier et à actualiser le règlement du Sénat pour le rendre plus lisible. Outre des modifications rédactionnelles à l'évidence pléthoriques concernant presque les deux tiers des articles de notre règlement, cette proposition de résolution vise trois objectifs. Elle vise tout d'abord à garantir la lisibilité et l'intelligibilité du règlement intérieur par la simplification et la clarification de la rédaction de certains articles, à l'instar de la règle de l'« entonnoir » ou encore de la procédure des propositions de par le rassemblement systématique des dispositions de nature semblable au sein d'articles ou de chapitres dédiés. Ainsi constate-t-on la création d'un chapitre spécifique aux organismes extraparlementaires ou la création d'un chapitre spécifique à l'organisation des travaux de commission. ensuite à simplifier et à assouplir notre ossature procédurale, en allégeant l'examen en séance publique- je pense notamment à la suppression, pour les procédures de nomination, des mécanismes de « double annonce » en séance publique en convertissant certaines obligations réglementaires annuelles en obligations pluriannuelles, à l'image de l'obligation de déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire, enfin, en introduisant une pointe de fluidité organisationnelle dans la planification des travaux par la conférence des présidents. Il s'agit en particulier de prévoir l'envoi, par le Premier ministre, des demandes d'inscription à l'ordre du jour prioritaire au plus tard la veille de la réunion de la conférence, ou de consacrer un délai pour la communication des sujets de contrôle. enfin à ajuster de façon bienvenue le cadre réglementaire à la réalité concrète des pratiques sénatoriales, en entérinant une certaine sénatoriale, à l'image des modalités de remplacement d'un membre du bureau ou d'un membre de commission hors session, ou encore de la possibilité pour une commission permanente de nommer plusieurs rapporteurs sur un texte. Il s'agit, en outre, de supprimer des dispositions jugées désuètes ou inappliquées. Je pense au scrutin public ordinaire en cas de doute sur la commission compétente, la référence aux procès-verbaux, à l'annonce du dépôt en séance des textes législatifs ou encore au dispositif des questions orales avec débat sur des sujets européens. Surtout, un signe ne trompe pas : cette révision du règlement s'opère à droit quasi constant et suivant une procédure de législation partielle en commission. Voilà bien une preuve, s'il fallait nous en convaincre, que notre outillage réglementaire ne manque pas de souplesse dans ses modalités d'exécution. Notre groupe fait tout de même valoir quelques réserves de fond. L'article 8 du règlement est modifié de telle sorte que ce sont désormais les « présidents » et non plus les « bureaux » des groupes politiques qui remettent au président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie pour siéger dans les commissions permanentes, sans préjudice- cela va sans dire -de la règle de proportionnalité. L'aspect discrétionnaire de la chose, renvoyant le souci de collégialité à une affaire de pratiques, semble, en cela, peu avisé. La modification de l'article 75 vise, quant à elle, à supprimer le temps de parole de « deux minutes et demie » prévu pour les questions d'actualité au Gouvernement, renvoyant sa fixation « temporelle » à la conférence des présidents. Nous doutons encore de l'opportunité d'une telle mesure. Nous aurions enfin souhaité apporter quelques utiles précisions sur le cadre applicable aux commissions d'enquête sénatoriales. L'affaire Benalla a révélé une pratique peu conforme à l'esprit transpartisan qui caractérise d'ordinaire une enquête sénatoriale. En effet, les membres de la commission des lois auraient sans doute apprécié de prendre connaissance, avant la levée de l'embargo médiatique, du rapport sur la base duquel ils étaient appelés à se prononcer. En dépit de ces quelques remarques, notre groupe apporte son soutien à cette révision. Merci

L'incertitude est grande concernant l'avenir du projet de réforme constitutionnelle du Président de la République et des projets de loi organique et ordinaire qui l'accompagnent. Si le retrait de l'inscription dans la Constitution d'un recul important concernant les droits du Parlement est un acquis, le fait de renvoyer ces modifications aux règlements des assemblées ne nous rassure pas. Le débat qui vient de se dérouler à l'Assemblée nationale, la réforme de son règlement votée- c'est une première ! -par la seule majorité, soulignent que les mauvais coups annoncés et portés durant un temps par Emmanuel Macron peuvent venir d'ailleurs. Cette réforme menée à l'Assemblée nationale confirme les violences faites au droit d'expression en matière tant de droit d'amendement que de temps de parole, là-bas, au Palais-Bourbon, comme ici, au Sénat. Limitation sans fin du temps de parole, rabougrissement du droit d'amendement, anéantissement de la possibilité de déposer des propositions alternatives et confinement de la séance publique au strict nécessaire : tout cela n'augure rien de bon pour l'avenir du pouvoir législatif. Ce qui fait la force des assemblées, c'est le débat, c'est la participation à l'élaboration de la loi, c'est le droit de modifier, voire de repousser, les propositions gouvernementales. Un Parlement qui ne débat plus, qui ne met pas en évidence la confrontation des idées, qui ne pousse plus la population à la réflexion en présentant des arguments bien étayés est un Parlement moribond Une démocratie qui perd son socle parlementaire est une démocratie vacillante, au bord du précipice. Pour tout vous dire, mes chers collègues, je ne comprends pas cette course à l'efficacité, chère au président Macron, mais relayée ici par la majorité. Les contradictions se multiplient d'ailleurs. Mercredi dernier, monsieur le président du Sénat, vous vous êtes inquiété, à juste titre, de la généralisation de la procédure accélérée pour l'examen des projets de loi et du recours aux ordonnances. Mais ne croyez-vous pas que la pression de l'exécutif est d'autant plus efficace que les assemblées se démunissent elles-mêmes de leur capacité d'exister, de peser, de faire respecter la Constitution ? Cet aveuglement est incompréhensible, à moins de supposer qu'il existe un accord sur le fond entre l'ensemble des partisans de l'ordre libéral qui exige l'affaiblissement des pouvoirs du Parlement, institution considérée comme un obstacle à l'expansion de l'économie mondialisée. N'exagérons rien ! Le Sénat qui a pourtant su montrer son utilité, sans doute du fait de son rapport étroit avec les préoccupations locales, peut se ressaisir et envoyer le signal que le Parlement dans notre République ne doit pas se désarmer. Or son arme, c'est le droit de s'opposer et celui de proposer

Il fut un temps, pas si lointain, où la majorité sénatoriale résistait à l'extension infinie des irrecevabilités. deux anciens présidents de la commission des finances et anciens rapporteurs généraux du budget, n'ont-ils pas proposé eux-mêmes d'abroger l'article 40 de la Constitution, ouvrant la voie à une plus grande capacité d'initiative financière du Parlement ? M. Hyest, rapporteur de la commission des lois sur le projet de révision constitutionnelle de 2008, ne s'est-il pas opposé avec ses collègues au transfert aux présidents des assemblées de la mise en oeuvre de l'article 41 de la Constitution, c'est-à-dire l'irrecevabilité dite « réglementaire » M. Hyest, pour défendre l'amendement visant à supprimer cette extension de l'irrecevabilité, déposé par la commission des lois du Sénat, déclarait dans son rapport : « Par ailleurs, on ne peut écarter que cette irrecevabilité, dès lors qu'elle serait soulevée à l'initiative des présidents des assemblées, soit appliquée lors du dépôt des amendements

La proposition du président Larcher fait entrer pleinement dans le règlement une conception particulièrement extensive de l'irrecevabilité, qui met en péril le droit d'amendement. En effet, les amendements seraient de plus en plus réduits à des commentaires de projets de loi et ne lors de la présentation de nos amendements, l'extension de la règle de l'entonnoir, qui, selon notre interprétation, pourrait devenir la règle dès la première lecture. Plusieurs présidents de groupe ont pourtant protesté contre ce développement des irrecevabilités qui tue le débat et désorganise la séance publique elle-même, comme nous le verrons tout à l'heure lors de l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique. J'espère qu'ils soutiendront notre démarche. Pourquoi se précipiter ainsi, monsieur le président ? Pourquoi graver dans le marbre du règlement des dispositions qui limitent encore nos pouvoirs de parlementaires ? J'évoquais l'incertitude du contexte. Pourquoi ne pas attendre confirmation ou infirmation de la réduction du nombre de parlementaires, autre grande menace contre nos assemblées, pour modifier un règlement qui devra tenir compte de cette éventuelle évolution ? Pourquoi cette précipitation ? Nous avons voulu cette discussion en séance publique, car l'heure est au redressement du Parlement et non à son avilissement. Nous sommes porteurs de propositions et nous souhaitons qu'elles soient examinées au grand jour et ne restent pas confinées à une salle de commission. En tout état de cause, si nos propositions de défense des droits du Parlement sont repoussées, nous ne voterons pas cette proposition de résolution,

l'activité parlementaire au Sénat. Il était nécessaire de faire évoluer un certain nombre de rédactions, comme l'a très bien dit notre président-rapporteur, Philippe Bas. Bas. Il est vrai que la réforme constitutionnelle, dont on peut penser qu'elle est menacée ou risque de ne jamais avoir lieu,

la procédure commune et généralisée. Il faudrait, pour le moins, que la conférence des présidents d'une assemblée puisse, dans un certain nombre de cas, s'opposer à ce que le Gouvernement impose la procédure d'urgence. d'urgence. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont vécu de très nombreuses années durant lesquelles la navette, la double lecture, était la règle, ce qui permettait de bien travailler et de peaufiner l'écriture des textes.

à ce temps perdu, à ce gâchis de travail parlementaire induit par le fait qu'une proposition de loi adoptée par une assemblée

de prévoir, comme l'avait suggéré un ancien président de la commission des lois, qu'une proposition de loi adoptée par une assemblée soit nécessairement examinée par l'autre assemblée dans l'année qui suit

J'aurai l'occasion de revenir lors du débat sur la question des commissions d'enquête. Il serait souhaitable, à la lumière d'une commission d'enquête récente,

même manière, il serait sage de revoir l'ordre d'examen des motions de procédure dans le cas d'une proposition de loi référendaire.

tendant à rédiger ainsi l'article 102 du règlement : « Les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions, à

tant pour les sénateurs que pour leurs collaborateurs qu'il fût clairement écrit que ceux-ci ont pour tâche d'assister les sénateurs dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exclusion de toute autre tâche. La parole est à M. Monsieur le président,

la procédure de législation en commission, le texte que nous examinons aujourd'hui est de faible portée politique. Il procède simplement du souhait du président du Sénat d'expurger notre règlement de références obsolètes, dont certaines sont des survivances de la III République.

C'était la grande époque du parlementarisme, qui a coïncidé avec le développement des progrès techniques ayant soutenu la croissance et la mondialisation au siècle dernier, que l'on pense à la construction de grands réseaux câblés à travers le monde ou à l'établissement du réseau de pneumatiques dans Paris. Leur développement ne s'est pas fait sans heurts. Ces histoires ne doivent pas être oubliées et sont porteuses de nombreuses leçons pour les nouvelles générations chargées de promouvoir les innovations futures. D'autres suppressions proposées, comme celle des questions orales avec débat remplacées par les débats d'initiative parlementaire, soulignent la capacité de notre Haute Assemblée à se rénover, servant souvent de modèle à l'Assemblée nationale. Bien que des marges d'évolution demeurent, les questions qui agitent aujourd'hui nos collègues députés ont depuis plus longtemps trouvé des réponses apaisées ici, qu'il s'agisse de la régulation du temps de parole en séance publique ou de l'allégement de la procédure parlementaire pour l'examen des réformes consensuelles. L'application de la procédure de législation en commission, la PLEC, à cette réforme du règlement en est le parfait exemple. Pour autant, et je l'évoquais à l'instant, certaines dispositions de notre règlement pourraient être remises en discussion sur le fond dans les mois à venir, comme le président du Sénat s'y était engagé lors de la préparation de la réforme institutionnelle. Nous allons le voir, certains de nos collègues souhaitent les aborder dès à présent. présent. Le président Bizet a par exemple exprimé sa volonté, au nom de la commission des affaires européennes, de renforcer le rôle d'alerte de cette dernière. Mais je pense, d'abord, aux procédures d'application des règles d'irrecevabilité. Elles contraignent fortement notre capacité d'action et ne sont pas suffisamment motivées, donc prévisibles. De façon générale, chaque fois que le Sénat cherche à se montrer vertueux dans la rationalisation de son activité parlementaire, il s'instaure une asymétrie de prérogatives entre lui et le Gouvernement, ou entre lui et l'Assemblée nationale. C'est le cas en matière de recevabilité des amendements, alors que la politique de l'Assemblée nationale en la matière donne à nos collègues de plus grandes marges de manoeuvre, quand bien même leurs initiatives sont ensuite censurées par le Conseil constitutionnel. Il n'en demeure pas moins que leurs propositions demeurent inscrites au compte rendu et peuvent nourrir les réflexions futures du législateur. C'est également le cas en matière de règles régissant le dépôt d'amendements, tandis que les sénateurs souffrent de délais plus contraints que le Gouvernement et tandis que la procédure accélérée est progressivement devenue la norme. Si, dans un premier temps, le parlementarisme rationalisé a fait ses preuves, je crois que, avec l'adaptation continue des pratiques parlementaires au nouveau cadre constitutionnel, il a échoué à améliorer la qualité de la loi, ce qui devrait pourtant être le premier des objectifs à rechercher. Des modifications du règlement pourraient être envisagées pour pallier ces limites, en faisant par exemple plus strictement observer le délai de réflexion de deux semaines entre l'examen en commission et l'examen en séance. Certains considèrent que le poids des lobbies et la porosité du Parlement à leur endroit est le premier responsable de cette dégradation législative. J'en fais une autre lecture. Je pense en effet que les réponses législatives aux problèmes concrets que rencontrent nos concitoyens pâtissent davantage des tentatives de contournement de règles d'irrecevabilité trop rigides et du rythme d'examen dorénavant extrêmement, voire trop, soutenu, amplifié depuis le passage au quinquennat. deux contraintes combinées dégradent considérablement notre capacité d'analyse et de formulation de solutions. Enfin, d'autres sujets pourraient être abordés à droit constitutionnel constant : le renforcement des droits des groupes minoritaires ou d'opposition notamment, avec l'introduction de la possibilité de leur attribuer le rapport lors de l'examen d'une proposition de loi déposée dans le cadre de leur ordre du jour réservé, comme je l'avais proposé. Enfin, tant l'affaire Fillon que l'évolution des rapports institutionnels, plaçant le Sénat en situation de « seul pouvoir constitutionnel non aligné », pour reprendre les mots du président Bas, ont ouvert la question des moyens humains mis à la disposition des parlementaires. Aux côtés de l'administration parlementaire, les collaborateurs dont nous nous entourons pourraient être ainsi mieux associés à nos travaux. Le groupe du RDSE porte ce sujet depuis longtemps. Nous avons conscience qu'il ne s'agit pas là du meilleur véhicule pour débattre de toutes ces questions : il n'a pas été conçu comme tel. Nous resterons donc dans une attitude d'écoute attentive aux propositions des uns et des autres, sans dévier de l'objectif initial. À moyen terme, si l'ajournement de la réforme institutionnelle écarte écarte la nécessité d'adapter nos règles de fonctionnement intérieures à l'évolution de notre loi fondamentale, il ne devrait pas retarder ces débats que beaucoup d'entre nous jugent vitaux pour l'avenir du parlementarisme. Le groupe du RDSE soutiendra cette proposition de résolution.

qu'il s'agisse de la suppression de la référence aux procès-verbaux qui n'existent plus depuis mars 2009 ou encore de celle des questions orales avec débat qui, elles non plus, n'existent plus depuis la même année et la création des débats d'initiative sénatoriale, il était temps de dépoussiérer notre règlement. Je salue donc la proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui par le président Larcher, car j'estime qu'elle est de bon sens. Cette proposition de résolution répond à des objectifs que je trouve particulièrement pertinents. Car l'application du triptyque visant à rendre plus lisible et plus facile d'accès le règlement, à simplifier et alléger certaines procédures, de même qu'à codifier des pratiques préexistantes et supprimer des dispositions obsolètes ou inappliquées, me semble d'une double utilité. Tout d'abord, il s'agit d'améliorer à droit « quasi constant » le travail quotidien du Sénat. C'est en quelque sorte notre « acte II » des réformes Larcher, traduisant la constance et la cohérence de la présente proposition de résolution résolution qui fait écho à celle de 2015 sur la réforme des méthodes de travail du Sénat, dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale. Par la suite, il s'agit de montrer l'exemple en n'appliquant rien de moins que des objectifs de valeur constitutionnelle d'accessibilité, d'intelligibilité et de clarté de notre règlement auprès de nos concitoyens. Je l'évoquais, la résolution de 2015 avait pour objectif de rendre le Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace. C'est également l'objet de la discussion de ce jour. Un Sénat plus présent, c'est un Sénat qui pérennise la mission de veille contre les surtranspositions, mission confiée à la commission des affaires européennes. Un Sénat plus moderne, c'est un Sénat qui adapte son règlement à la mise en place du scrutin public électronique, prévue à compter du 1 octobre prochain. Un Sénat plus efficace, c'est un Sénat qui allège la séance publique, facilite la planification des travaux par la conférence des présidents, ou encore intègre des règles relevant de la pratique. Cet utile effort de clarification supprime des dispositions qui recueillaient un large et rare consensus politique quant à leur obsolescence, qu'il s'agisse des délégations de vote « par télégramme » ou des pétitions réunies au sein d'un « feuilleton » qui n'est plus publié depuis de nombreuses années. Comment, par ailleurs, ne pas soutenir la suppression d'une mesure découverte lors de l'examen de cette proposition de résolution, selon laquelle, lors des scrutins publics, les secrétaires doivent se tenir dans le couloir droit de l'hémicycle pour les votes « pour » et dans le couloir gauche pour les votes « contre » ? De telles dispositions sont anachroniques et leur suppression est la bienvenue. Je tiens également à saluer le travail exemplaire de la commission des lois, dont le rapporteur a soutenu les propositions de nombreux collègues- ils ont vu leurs amendements adoptés et intégrés accueillant avec bienveillance les contributions diverses à l'amélioration et la modernisation de notre charte commune. Nous pouvons être fiers de l'exemplarité avec laquelle se sont tenus des échanges inscrits dans la tradition du pluralisme sénatorial et ne donnant pas lieu à de bruyantes et contre-productives postures. Je tiens à me féliciter de la méthode, avec une consultation constructive de tous les groupes politiques en amont, ainsi que des échanges nourris entre le rapporteur et l'ensemble des présidents de groupe et de commission pour s'assurer de l'absence d'objections à cette révision et recueillir leurs suggestions bienvenues. Cette résolution sort enrichie de débats constructifs, qu'il s'agisse des droits attribués aux groupes au début de chaque année, des précisions quant au contrôle de recevabilité financière ou sociale, mais également des conditions de travail de nos collaborateurs, avec la pérennisation d'une cellule d'écoute et d'accueil pour assurer un travail parlementaire juste et équilibré. Faire évoluer le Sénat et son fonctionnement au quotidien, c'est améliorer son image et participer d'une plus grande transparence de son fonctionnement et de son apport non négligeable au travail parlementaire. Vous le savez, notre institution est parfois la mal-aimée de la République, car incomprise, critiquée car à l'écart de la politique médiatique, celle-là même qui se trouve être à bout de souffle et ne convient plus à nos concitoyens. Loin d'une institution obscure, cette proposition de résolution donne les moyens de faciliter et simplifier le travail parlementaire. Loin d'une institution sclérosée, cette proposition de résolution illustre une institution qui se donne les moyens de la transparence et de la modernisation. D'ailleurs, je constate que plusieurs innovations issues de la « réforme Larcher » de 2015 ont inspiré nos collègues de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse du contrôle du respect du domaine de la loi et du règlement, de la législation en commission. Le Sénat peut être assurément fier de ses initiatives qui ont permis d'améliorer nos procédures tout en respectant les droits des groupes minoritaires et d'opposition. Si, dans un second temps, des modifications de fond plus substantielles sont envisageables, en écho aux réformes institutionnelles à venir, cette proposition de résolution traduit un exercice consensuel et pragmatique de remise en cause constructive et d'améliorations textuelles qui rendront, j'en suis convaincu, le travail parlementaire encore plus efficace. Le groupe Union Centriste votera assurément en faveur de ce texte. La parole

collègues, la sédimentation de ses dispositions au fil des années- pour ne pas dire des Républiques -rend souvent notre règlement difficile d'accès, se traduisant par des règles éparses, des mesures parfois totalement obsolètes ou encore des procédures inutilement complexes. Texte très technique, cette proposition de résolution modifie une centaine d'articles de notre règlement- soit presque les deux tiers du nombre total d'articles qu'il contient -et tend à créer une vingtaine d'articles nouveaux. Cette proposition de résolution répond à un triple objectif, qui se caractérise par son aspect à la fois simple et pragmatique : clarifier, simplifier et codifier. Clarifier, tout d'abord, en rendant plus lisible et plus facile d'accès le règlement du Sénat ; simplifier, ensuite, en allégeant certaines procédures en séance publique, en rendant pluriannuelles certaines obligations annuelles ou encore en facilitant la planification des travaux par la conférence des présidents codifier, enfin, des pratiques préexistantes ou résultant de la conférence des présidents, mais également supprimer des dispositions obsolètes ou inappliquées. à saluer, à cette tribune, le travail du rapporteur et président de la commission des lois, notre collègue Philippe Bas, qui, pleinement respectueux de la démarche lancée par le président Gérard Larcher, a tenu à en conserver l'esprit et n'a donc pu retenir les amendements qui tendaient à proposer des innovations ou des évolutions trop éloignées de nos méthodes de fonctionnement actuelles. Dans ce cadre, je me félicite de ce que la commission ait prévu plus explicitement l'intervention de la conférence des présidents concernant les droits attribués aux groupes au début de chaque année, pour lui permettre d'examiner avec souplesse leur situation, notamment si des modifications importantes intervenaient en cours d'année parlementaire. Je me réjouis également que la commission ait consacré et précisé le rôle des présidents des commissions des finances et des affaires sociales dans le contrôle de recevabilité financière ou sociale, et qu'elle ait intégré la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la tenue de jours supplémentaires de séance sur demande du Gouvernement. Enfin, je voudrais mettre l'accent sur l'utilité de deux autres dispositions : l'adaptation de notre règlement à la mise en place du scrutin public électronique, prévue à compter du 1 octobre 2019, d'une part, et la pérennisation de la mission de veille contre les surtranspositions confiée à la commission des affaires européennes, d'autre part. Mes chers collègues, cette proposition de résolution révisant le règlement du Sénat est à droit « quasi constant » : elle procède soit par des modifications de pure forme, soit par des reformulations de fond, soit encore par des harmonisations de régimes ou par l'explicitation de pratiques parlementaires ou de jurisprudences Le groupe Les Indépendants approuve pleinement cet effort utile de clarification et de dépoussiérage de nos règles communes, dont l'initiative revient au président Larcher et qui a bénéficié en commission des apports et des amendements des différents groupes parlementaires.

Monsieur le président, mes chers collègues, la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui est le fruit d'un effort de concertation effectué bien en amont. Ce travail a impliqué l'ensemble des groupes politiques de notre Haute Assemblée. De prime abord, les changements apportés par cette proposition de résolution peuvent sembler considérables ou substantiels, dès lors qu'elle tend à modifier quasiment les deux tiers des articles du règlement du Sénat et à introduire une vingtaine de nouveaux articles. Néanmoins, en dépit de son volume, le texte que nous examinons aujourd'hui s'articule autour d'un objectif distinct : celui de permettre à notre règlement de gagner en lisibilité et en cohérence. En effet, en l'état, la sédimentation successive des dispositions, année par année, a rendu ce dernier difficile d'accès, voire quelque peu ésotérique. À titre d'exemple, les nombreuses règles dispersées en plusieurs chapitres contribuent à en complexifier la compréhension, ce qui n'est jamais bon. C'est notamment le cas des règles relatives à la composition et à la procédure de désignation du Bureau à la proportionnelle, actuellement dispersées entre les articles 2, 3 et 6. Notre règlement comprend, en outre, un certain nombre de dispositions dont l'obsolescence n'est plus à prouver. Concernant les délégations de vote, en son article 64, il précise ainsi : « En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sous réserve de confirmation immédiate dans les formes prévues ci-dessus. ci-dessus. En ce cas, la délégation cesse d'avoir effet à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception du télégramme si, dans ce délai, une lettre de confirmation signée du délégant n'a pas été reçue par le Président du Sénat. On voit sans difficulté le caractère périmé du texte. En son article 89, le règlement dispose qu'un « feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres du Sénat faire appel au souvenir des plus anciens pour trouver trace d'un tel « feuilleton », qui n'a pas été publié au sein de notre assemblée depuis bien longtemps. Concernant les scrutins publics enfin, en son article 56, le règlement actuel prévoit que « les sénateurs votant " pour " remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite de l'hémicycle un bulletin blanc » et que « les sénateurs votant " contre " remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche de l'hémicycle un bulletin bleu

! La présente proposition de résolution vise ainsi à clarifier et actualiser le contenu du règlement, afin de concourir à la clarté de la norme parlementaire et d'assurer une meilleure adéquation entre celle-ci et le travail parlementaire tel qu'il est effectué. Nous accueillons donc favorablement cette proposition de résolution, et ce d'autant plus que la révision proposée se fait- cela a été dit -« à droit " quasi constant ", c'est-à-dire en procédant soit par modifications de pure forme pure forme (déplacements, modernisations de style), soit par reformulations de fond (recodifications, clarifications, simplifications), soit encore par des harmonisations de régimes ou l'explicitation de pratiques parlementaires ou de jurisprudences constitutionnelles En effet, les changements ou ajouts opérés ne modifient pas la substance de la procédure parlementaire devant le Sénat. Ces derniers se limitent à reconnaître des usages devenus coutumiers ainsi qu'à clarifier et mettre à jour le règlement, notamment en élaguant des dispositifs devenus manifestement obsolètes. C'est ainsi le cas des articles relatifs aux délégations de vote par télégramme, qui sont remplacés par des dispositions sur le recours aux outils électroniques. Cette démarche de simplification est donc la bienvenue et je remercie le président Larcher de cet effort salutaire de clarification de nos règles communes, qui est présenté comme une première étape avant d'envisager, dans un second temps- nous l'espérons tout du moins -, des modifications de fond bien plus substantielles. Je pense que les réformes institutionnelles qui nous occuperont bientôt permettront d'évoquer ces questions et de prolonger nos efforts afin de rendre le travail parlementaire encore plus efficace. Je ne doute pas que nous aurons, à ce titre, de nombreuses propositions à formuler afin de consolider les outils de contrôle de l'action du Gouvernement et de veiller à ce que les politiques publiques répondent aux attentes de nos concitoyens et de nos territoires. Pour toutes ces raisons, je voterai donc en faveur de cette proposition de résolution.

prendre acte des dispositions de clarification et d'actualisation de notre règlement, introduites par le président Gérard Larcher et parfaites par la commission des lois du Sénat. Comme le président-rapporteur Philippe Bas vient de nous le rappeler, il « s'est [ ...] assuré que cette révision du règlement se fasse bien [ ...] à droit " quasi constant ", c'est-à-dire en procédant soit par modifications de pure forme pure forme (déplacements, modernisations de style), soit par reformulations de fond (recodifications, clarifications, simplifications), soit encore par des harmonisations de régimes ou l'explicitation de pratiques parlementaires ou de jurisprudences constitutionnelles Un objectif qui n'est pas sans rappeler, dans un autre registre, celui de la mission Balai, d'après le bien nommé bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles, de notre collègue Vincent Delahaye. Hasard de calendrier, à l'Assemblée nationale, on débattait également, de façon plus spectaculaire qu'ici, il y a quelques jours, avec des centaines d'amendements déposés, d'une proposition de résolution tendant à modifier le règlement de celle-ci. tout l'intérêt d'un Parlement bicaméral pour le bon fonctionnement de nos institutions, et toute l'importance du travail sénatorial pour l'apaisement du débat public. Relevons tout de même un élément intéressant de notre débat, en commission la semaine dernière et en séance publique aujourd'hui : le présent texte laisse percevoir, dans cet hémicycle et dans l'autre chambre parlementaire, un vif débat que nous serons amenés à avoir dans le cadre d'une éventuelle future révision constitutionnelle. J'identifie trois principaux enjeux, qui se manifestent par de petits amendements ou de courtes introductions dans le règlement, mais qui semblent illustrer une tendance profonde au sein de notre institution. Le premier enjeu est celui de la place et du rôle des collaborateurs de groupe et collaborateurs parlementaires, avec les amendements portés par un certain nombre de nos collègues. La création récente d'une instance de dialogue social entre sénateurs et collaborateurs ainsi que les premières élections professionnelles à la fin du mois semblent annoncer une affirmation du rôle des collaborateurs dans cette maison. La répartition factuelle du travail entre ceux-ci et les administrateurs doit être l'occasion non pas d'une forme de concurrence entre ces deux catégories d'interlocuteurs du sénateur, mais d'une réaffirmation de la place centrale du sénateur. Le deuxième enjeu que j'identifie est celui de la place des groupes minoritaires dans les débats et travaux parlementaires. Le droit de ces groupes est un fondement incontournable du bon fonctionnement et de la vivacité de notre démocratie. Le troisième enjeu est celui du droit d'amendement et la question de la recevabilité financière. J'ai vu passer, en particulier, des amendements visant à pousser la commission des finances à publier des avis motivés pour chaque décision de rejet pour irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. Compte tenu du nombre d'amendements déposés par texte et de l'état de nos finances publiques, nous pourrions plutôt attendre des parlementaires que nous sommes, dans l'exposé des motifs, une meilleure évaluation des amendements et une justification de leur recevabilité ou soutenabilité du point de vue des finances publiques. Cette question pourrait être posée à l'occasion d'une révision constitutionnelle. En tout état de cause et de toute évidence, je suivrai l'avis du président et rapporteur Philippe Bas sur ce nouveau règlement. La parole

D'autant qu'elle ouvre la possibilité du dépôt ultérieur d'une proposition de résolution complémentaire comprenant des modifications de fond, après une nouvelle concertation avec les représentants des groupes. La résolution de ce jour et la résolution ultérieure, déjà entrevue par le président Larcher, mettront notre procédure parlementaire définitivement à l'abri d'une révision institutionnelle totalement imprévisible dans le temps et dans ses formes. Je place ma brève intervention dans cette optique, en soulevant deux points qui nécessitent un débat de fond. en premier lieu, de deux motifs d'irrecevabilité de nos amendements. L'article 45, alinéa 1, de la Constitution, prévoit que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Cette disposition est reprise aux articles 28 et 48, alinéa 3, du règlement du Sénat. Elle a même fait l'objet d'un vade-mecum, distribué par les services de notre assemblée. Il ressort de ces dispositions qu'il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur ces cas d'irrecevabilité, appelés « cavaliers ». L'appréciation du lien d'un amendement avec le texte étant d'ordre politique, elle doit nécessairement faire l'objet d'une réelle discussion en commission. Pourtant, il semble que cela ne soit pas toujours le cas. Le plus souvent, le sort de l'amendement relève de la prédestination, décidée par les services et le président de la commission. Si l'amendement qui portait de douze à quatorze semaines le délai de l'IVG avait été soumis à la discussion de la commission, celle-ci se serait rendu compte qu'il se rattachait à la loi de façon très ténue et que son objet nécessitait un débat de fond. En conséquence, elle l'aurait fait passer à la trappe au nom de l'article 45, ce qui nous aurait évité un psychodrame en séance publique. Mais le cas le plus préoccupant concerne l'article 40 de la Constitution, selon lequel « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Les articles 28 et 45 du règlement du Sénat confient le contrôle de la recevabilité financière à la commission des finances. Ce principe est réaffirmé par la présente proposition de résolution. Comme précédemment, il ressort de ces dispositions que la recevabilité financière des amendements doit être discutée en commission, c'est-à-dire présentée aux commissaires avec le motif d'irrecevabilité. Mais, en pratique, tout est décidé par les administrateurs et le président de la commission. Les amendements sont proprement « exécutés » au coin du bois ! Personne n'en entend plus parler puisqu'ils disparaissent de la circulation : ils deviennent les « invisibles du Sénat Pourtant, la discussion en commission de la recevabilité financière des amendements permettrait de limiter l'extension démesurée de l'article 40 de la Constitution par le Sénat. Car l'Assemblée nationale, elle, ne transforme pas l'article 45 en robe de bure et l'article 40 en cilice En deuxième lieu, je veux évoquer le contrôle des ordonnances. Aux termes de l'article 38 de la Constitution, « les ordonnances « deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation le Sénat est une assemblée permanente, tous les gouvernements ont pris l'habitude de déposer les projets de loi de ratification sur le bureau de notre assemblée. Les ordonnances étant d'application immédiate, le Gouvernement a ainsi tout le temps devant lui pour faire procéder à la ratification, le plus souvent au moyen d'articles figurant dans des projets de loi à portée générale comme la loi Pacte, ou même, au dernier moment, par voie d'amendement. Le Parlement, dans ces conditions, n'a ni le temps ni les moyens de contrôler l'usage que le Gouvernement a fait de la délégation de son pouvoir législatif. Il arrive même qu'il n'y ait aucun contrôle du tout, car peu de lois de ratification sont inscrites à l'ordre du jour ès qualités. À l'issue de la session 2017-2018, il y avait ainsi un « stock » de 38 textes en instance. À l'évidence, il existe là une carence du contrôle de l'action gouvernementale, que nos semaines prévues à cet effet ne comblent pas. Une concertation exigeante est donc à mener avec le Gouvernement pour permettre un contrôle continu des ordonnances, lesquelles devraient d'ailleurs être cantonnées à des sujets techniques, ce qui est loin d'être le cas actuellement. La parole

qui est évidemment limité dans son ambition et sa portée. En effet, il s'agit d'assurer la lisibilité et la maniabilité de notre

d'accès pour le justiciable. On a beau dire que nul n'est censé ignorer la loi, la vérité pratique, c'est que la loi est généralement ignorée, tout simplement parce que la loi d'aujourd'hui est devenue obèse et boursouflée.

Et je prends en compte non pas les modifications d'articles, mais seulement l'ajout de nouveaux articles par amendement. Notre pouvoir d'amendement s'exerce donc heureusement pleinement. Il faut donc garder à l'esprit la dimension réelle

à débattre de bien d'autres sujets que vous avez, mes chers collègues, abordés à la tribune. Je vous propose de le faire à l'occasion de l'appel des amendements qui en feront l'objet.

car il nous paraît étonnant, voire improbable, de discuter des conditions du renouvellement des plus hautes instances du Sénat au sein de la seule commission des lois. Je me félicite d'ailleurs du nombre de parlementaires qui sont aujourd'hui présents pour débattre de ce texte. Vous allez me répondre, monsieur le président Bas, que nous sommes à droit constant ou quasi constant. Mais une telle affirmation ne tient pas compte de la volonté des parlementaires et des groupes de faire débattre de propositions par l'ensemble du Sénat, de déposer des amendements et de pouvoir les voter, quelle que soit

Nous considérons que le fait majoritaire s'applique de manière particulièrement excessive ici, comme d'ailleurs à l'Assemblée nationale. La composition du bureau du Sénat est, à ce titre, caractéristique d'une répartition faite au détriment de l'opposition, en particulier des groupes minoritaires et des petits groupes. Faut-il rappeler qu'un groupe, fût-il faible en nombre, doit affronter l'ensemble de la vie parlementaire- et je crois que mon groupe en est un bon exemple. est particulièrement vrai pour l'activité législative et en séance publique. Il nous paraît donc légitime que chaque groupe qui le souhaite ait droit à un poste de vice-président, fonction dont on connaît l'importance dans la vie démocratique de notre assemblée. Nous proposons que chaque groupe dispose d'un tel poste ou, si le groupe peut y prétendre, d'un poste de questeur, libérant ainsi un poste de vice-président. Il s'agit, pour notre groupe, non pas

! Par conséquent, la commission est, pour ce type de procédure, ouverte à l'ensemble les sénateurs.

des fonctions de responsabilité, telles que celles de vice-président et de questeur, se fait à la proportionnelle des groupes, et dépend donc des effectifs de ceux-ci. Cette règle n'est pas nouvelle, je comprends que certains groupes, dont le vôtre, puissent avoir à en souffrir. Néanmoins, on ne peut pas changer la règle en fonction des circonstances. C'est la raison pour laquelle nous avons donné un avis défavorable l'autre raison étant bien sûr qu'il s'agit d'un changement de règles de fond, qui aurait d'ailleurs un impact sur la représentation des autres groupes dans les fonctions de vice-président ou de questeur.

Demander à ce que tout groupe ait un vice-président ou un questeur, sauf à dire qu'il y aura vingt vice-présidents et dix questeurs, me semble quelque peu difficile, puisque, dans le même temps, vous êtes les premiers à dire- et c'est bien normal -que notre Haute Assemblée ne doit pas augmenter ses dépenses de fonctionnement.

Le bureau du Sénat est une instance essentielle, vous le savez, mes chers collègues. Des questions aussi diverses que le budget du Sénat, ses finances, sa communication ou des instructions générales concernant son fonctionnement concret y sont notamment abordées. Un compte rendu succinct existe. Nous pensons qu'il devrait être détaillé et accessible au plus grand nombre. Nous estimons, en revanche, que les délibérations devraient être bien sûr exclues, comme dans le cadre des incompatibilités ou des saisines de justice consécutives à une procédure de commission d'enquête. Sur ces Sur ces derniers points, nous estimons que la procédure du vote à main levée devrait être généralisée, afin de permettre une plus grande transparence des votes au sein même du Bureau.

Cette mesure, sans être une révolution, peut contribuer à cet effort de publicité, de clarté de notre fonctionnement. Selon nous, il serait judicieux de le faire savoir. Quel est l'avis

M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit de préciser dans le règlement ce qui est déjà un fait, à savoir que les réunions des commissions donnent lieu à un compte rendu analytique. En effet, très souvent maintenant, vous le savez, ce sont les fonctionnaires du compte rendu analytique qui viennent en commission rédiger un compte rendu particulièrement précieux.

d'avoir ici un compte rendu intégral et un compte rendu analytique que nous pouvons retrouver chaque jour et qui est, j'y insiste, extrêmement précieux pour la compréhension de nos travaux. Puisque c'est le cas,

Je suis toujours ravi d'échanger avec le président Sueur sur des questions de sémantique. Actuellement, le compte rendu est détaillé : toute la portée de l'amendement de notre collègue est de dire que le compte rendu détaillé est en réalité un compte rendu analytique. Si l'on veut uniformiser, on pourrait dire que le compte rendu de nos débats est détaillé, comme celui des commissions, ou que le compte rendu de nos commissions est analytique, comme celui de nos débats ... En réalité, pour ce qui me concerne, je ne sais plus faire la différence entre un compte rendu détaillé et un compte rendu analytique. Je dois dire que les rédacteurs de ces comptes rendus ne la font pas non plus. Si bien que je crois, cher président Sueur, qu'il n'y a pas de désaccord de fond entre nous ; mais je ne sais pas,

reprendre chacun des articles mentionnant un compte rendu soit détaillé, soit analytique, pour ajuster toutes les rédactions. Or votre amendement porte sur les seuls comptes rendus détaillés

5 est-il maintenu ? Ma bonne volonté est extrême, mais je crois très important de défendre l'existence, la pertinence, l'utilité et la nécessité du compte rendu analytique. Par conséquent, je ne retire pas cet amendement.

de la Chambre des représentants de la République de Chypre, conduite par son président, M. Giórgos Lillíkas. Elle est accompagnée par notre collègue Nelly Tocqueville, présidente du groupe d'amitié France-Chypre. La délégation est à Paris pour évoquer tant la partition de l'île que les questions énergétiques. Elle s'entretiendra avec nos collègues Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, et Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes. Le Sénat entretient d'excellentes relations avec la Chambre des représentants chypriote, et la France en est un partenaire étroit, comme en témoignent les contacts fréquents entre nos deux pays. Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, la plus cordiale bienvenue et un fructueux séjour à nos homologues de la Chambre des représentants de Chypre.

Il n'est pas question pour moi de remettre en cause la qualité des administrateurs des commissions ou des administrateurs en général. Je dis simplement que nous nous trouvons dans la plus parfaite contradiction, dans

Nous avons toutes les raisons, en effet, d'exprimer notre reconnaissance pour le travail que ces derniers accomplissent à nos côtés. C'est nous qui définissons, en fonction de ce que nous sommes et de ce qu'est notre besoin, le travail de nos collaborateurs. Certains, d'ailleurs ne participent aucunement au travail législatif ; ils nous assistent dans nos relations avec les forces vives et les élus de nos circonscriptions ; d'autres prennent en charge l'organisation de notre agenda, les questions d'actualité, les questions écrites ; enfin, certains d'entre eux nous assistent dans l'élaboration de nos amendements. Une minorité d'assistants parlementaires peuvent également nous apporter leur concours lorsque nous sommes rapporteurs d'un texte et ils le font généralement- vous avez raison de le souligner, monsieur Karoutchi -avec beaucoup d'efficacité, ce que nous avons toutes raisons de louer.

où nous faisons notre rapport s'assoie à nos côtés un assistant parlementaire, plutôt qu'un administrateur, pour nous éclairer sur le sens de la réponse qui nous a été préparée en vue d'émettre un avis favorable ou défavorable à un amendement examiné en commission.

tel un témoin muet, mais qui sera ainsi parfaitement informé de ce qui se passe dans la préparation du rapport, d'être présent- non

dernier m'a autorisé à vous dire qu'il prenait l'engagement d'ouvrir une concertation sur les bases que je viens de définir et sur lesquelles il m'a donné son accord. Cela nous permettrait d'avancer, mais dans

demande de bien vouloir retirer votre amendement, fort de l'engagement que je prends devant vous, au nom du président du Sénat, d'ouvrir la concertation sur le sujet que vous avez abordé et pour lequel je suis davantage d'accord avec le propos que vous venez de tenir publiquement qu'avec le texte même de l'amendement. De mon point de vue, celui-ci ne reflète pas exactement ce que vous nous avez dit.

de collaborateurs, collaborateurs de groupes et assistants parlementaires, qui peuvent être autorisés par le président de chaque commission

différentes associations de nos collaborateurs ainsi que les représentants des administrateurs pour trouver le bon réglage. Mes chers collègues, l'objectif

que la confiance que je fais au président de la commission des lois et au président du Sénat n'a plus lieu d'être. Je le dis de la manière la plus claire. J'accepte de retirer mon amendement, à la seule condition que la confiance ne soit pas rompue.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

les membres du groupe socialiste et républicain ont voté votre amendement lors de la réunion de commission qui vient d'avoir lieu. Toutefois, comme vous le savez aussi, nous avons assorti notre approbation de deux points déjà largement

La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

bien écoutés, les uns et les autres. Je voudrais répondre à la préoccupation de la confiance. Vouloir que le Bureau soit saisi, rédiger un texte qui fait obligation au Bureau, en ce qu'il utilise l'indicatif présent, de prendre de nouvelles dispositions, c'est déjà un gage de confiance.

notre règlement, le président du Sénat a effectivement procédé à des concertations. Les concertations ne doivent pas être de la procrastination. Elles doivent être utiles et permettre de trouver les solutions en y incorporant

aux collaborateurs des auteurs de propositions de loi d'être présents aux auditions, pour être pleinement et en temps réel informés du travail de leur sénateur sur une proposition ou un projet de loi, et d'être également présents

au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que l'on puisse déroger à cette règle, même si, encore une fois, je suis extrêmement soucieux qu'un maximum de rapports puissent être

J'ai participé longuement à des débats à l'Assemblée nationale. Je me souviens que Georges Hage présentait le budget des sports. Il était extraordinaire. Il rapportait toujours

au titre de l'article 40 de la Constitution soit émise par un avis écrit et suffisamment motivé. Quel est l'avis

de légitimer davantage les irrecevabilités financières, qui sont un irritant pour le travail parlementaire, en particulier pour les auteurs des amendements concernés. Je crois

demande au président de la commission des finances. Comme président de commission, je trouve que cela ralentirait considérablement notre travail parlementaire. Imaginez que nous interrompions toutes les séances de commission, déjà extrêmement chargées, pour aller faire avaliser

nous touchons au coeur du débat sur le rôle du Parlement et sa place dans notre démocratie. J'avoue ne pas bien comprendre- je l'ai déjà indiqué -l'obsession de la réduction de ce droit d'expression. Cette obsession d'un parlementarisme rationalisé masque mal une volonté d'étouffer le débat pluraliste

d'étude ... Le temps de parole ou le droit d'amendement ont bon dos pour expliquer la surcharge de travail ! Le débat réellement public est une des clés de la démocratie. C'est l'essence même du Parlement que de permettre la confrontation des idées. L'expérience montre déjà que le débat en commission ne peut pas suppléer la séance publique ; j'en veux pour preuve ce qui s'est passé cet après-midi. Elle montre aussi que, lorsque le Parlement ne joue plus son rôle, en raison soit de sa représentativité fragile et insuffisante, soit de son manque de pouvoir, le débat a lieu ailleurs, et la colère peut rapidement monter. monter. Nous estimons donc que les pouvoirs et majorités successifs ayant corseté le débat parlementaire portent une responsabilité directe dans la crise politique et institutionnelle actuelle. C'est une course

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement n'a rien de révolutionnaire : il vise à revenir à la situation qui prévalait voilà quelques années en matière de temps de parole de référence, en dehors des discussions générales et débats. Deux minutes et demie pour effectuer un rappel au règlement, défendre un amendement ou expliquer un vote sur article peut se révéler tout à fait insuffisant. Cette restriction systématique du droit d'expression relève d'une critique du débat, jugé en soi inutile ou superfétatoire. Nous vivons dans une société du zapping, marquée par l'accélération de l'information liée aux réseaux sociaux. Le Parlement est l'endroit où une résistance à cette évolution peut s'organiser. C'est ce que nous proposons de faire au travers du vote de cet amendement. Quel

autres activités qu'il lui est loisible d'avoir en dehors des heures de service ... Cela prend quinze secondes ! Moi aussi, j'aime le Parlement, et même si mon expérience de celui-ci est est moins large que la sienne, je parviens à comprendre toute la saveur qu'il retire de ces phrases sacramentelles que les présidentes et présidents prononcent à la fin des séances.

il faut réunir plus de 185 signatures de parlementaires pour déposer la proposition de loi référendaire. Ensuite, il est nécessaire de réunir plus de 4,7 millions de signatures de nos concitoyens pour franchir la seconde étape, qui est sans nul doute la plus difficile, car nous constatons aujourd'hui que les dispositions législatives sont imparfaites du point de vue du citoyen : publication des noms- elle inquiète et dissuade -, absence de comptage- elle ne permet pas de mesurer la mobilisation -, absence de moyens d'information audiovisuels ou à l'échelon local ... Enfin, une fois les signatures recueillies, la proposition de loi référendaire est de nouveau soumise au Parlement. le cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution dispose : « Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. » Il faut donc créer les conditions pour qu'une assemblée puisse majoritairement refuser d'examiner une telle proposition ! Or le règlement du Sénat, tel qu'il est rédigé, autorise un groupe politique, même minoritaire, à déposer une motion portant irrecevabilité ou question préalable. Que

dans le cas de la mise en oeuvre de l'article 11 de la Constitution, être déposée et défendue préalablement à toute autre motion, ce qui permettrait au Sénat d'exprimer majoritairement son refus d'examiner la proposition de loi référendaire. Enfin, et c'est un point important, il apparaît nécessaire de modifier le règlement du Sénat pour qu'un renvoi en commission soit pleinement effectif, même lorsque le Gouvernement inscrit à l'ordre du jour la proposition de loi, en supprimant l'obligation faite à la commission de présenter dans ce cas son rapport lors de la même séance.

d'inscrire l'examen de cette question à son ordre du jour prioritaire, les règles applicables sont très claires

qui empêchent la correcte application sur ce point de la révision constitutionnelle de 2008. Je reconnais toutefois le très grand intérêt du travail qui a été

Le Conseil constitutionnel a certainement des choses à dire sur cette question, et puisque le règlement du Sénat lui est nécessairement transmis, rien ne l'empêcherait de se prononcer sur ce point pour donner sa pleine portée aux dispositions de la Constitution. Quoi qu'il en soit, j'émets

à Mme Laurence Cohen. Nous l'avons déjà souligné, le développement anarchique des irrecevabilités mises en oeuvre au nom des articles 40, 41 et 45 de la Constitution

Peut-on parler de débat lorsque les partis sont écartés de celui-ci ? Déposer un amendement, obtenir le label de recevabilité, le faire examiner en commission ou en séance publique devient un véritable parcours du combattant Pis, nous avons bien souvent l'impression que la décision de recevabilité d'un amendement relève de la loterie et du bon vouloir de telle ou telle personne. D'ailleurs, qui décide vraiment de la recevabilité ? Cela s'apparente bien souvent à un mystère

aux finances publiques, la LOLF, qui a fini de réduire le débat budgétaire à néant, ou presque. J'ajoute, enfin, que cette disposition permettrait d'éviter la confusion actuelle, née des déclarations d'irrecevabilité intervenant en cours de discussion, empêche les groupes et parlementaires d'avoir une vision claire du débat. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement de bon sens- démocratique, devrais-je dire. L'amendement n° 28, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous proposons que toutes les catégories d'irrecevabilité émises par la commission des finances fassent l'objet d'un avis écrit et motivé de manière non tautologique.

C'est là un point très important, car nous sommes contre la possibilité laissée à la commission des finances de se saisir de tout amendement sur n'importe quel texte passant devant n'importe quelle commission. Ici, nous sommes cohérents avec notre amendement à l'article 17 du règlement, par lequel nous proposions que la commission des finances soit saisie des seuls amendements que lui transmet le président de la commission saisie au fond. Nous proposons, enfin, qu'aucune irrecevabilité ne soit accordée de façon tacite en cas de non-réponse

une contrainte constitutionnelle, laquelle a donné lieu à une abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il serait vain de vouloir faire mettre en discussion des amendements irrecevables, car le Conseil constitutionnel se saisit toujours d'office, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin que la saisine des députés ou des sénateurs ne mentionne le caractère irrecevable d'un certain nombre d'amendements éventuellement adoptés. Par conséquent, tous ces efforts, que je comprends très bien et qui sont d'ailleurs appuyés sur une réflexion technique approfondie, me

M. André Reichardt, pour explication de vote.

en interrogeant la commission des finances, qui était précisément en train de travailler sur ce dossier et qui a élaboré assez récemment une sorte

vote. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mon explication vaut pour l'article 40, mais aussi pour l'article 45

est à M. Fabien Gay. Monsieur le président de la commission des lois, les dispositions de notre amendement ne relèvent pas de la seule précision sémantique. Le règlement actuel fait une distinction entre l'étape où l'amendement doit avoir un lien effectif- au cours de la seconde lecture -, et un lien direct ou même indirect- au cours de la première lecture. La rédaction actuelle prévoit que « les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou- et j'insiste sur ce -s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion ». La nouvelle rédaction remplace ce « ou » par un « et ». Ainsi les amendements doivent-ils s'appliquer effectivement au texte et avoir un lien direct ou indirect

Ainsi sommes-nous portés à estimer que la volonté de l'auteur est d'appliquer la règle de l'autonomie, dès la première lecture, en obligeant, de toute façon, à un lien effectif. convenez, mes chers collègues, qu'il existerait une contradiction manifeste entre le fait d'exiger, dès la première lecture, ce lien effectif, tout en autorisant un lien indirect. Devant cette confusion possible et le risque d'ouvrir la voie à une réduction drastique du droit d'amendement, nous proposons d'en rester à la rédaction actuelle du règlement. Sinon, vous en conviendrez, monsieur le président, nous sortons du droit constant, et même du droit quasi quasi constant. Nous attendons avec intérêt vos explications en ce domaine. Quel

Jean-François Longeot. Cet amendement vise à préciser les amendements recevables, ou non, au titre de l'article 45 de la Constitution, lequel mentionne clairement que les amendements doivent avoir un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Au travers de cet amendement, nous entendons préciser que les dispositions introduites à l'Assemblée nationale peuvent être amendées ou précisées au Sénat. L'interprétation de l'article 45 de la Constitution doit être en faveur de l'initiative parlementaire et du pouvoir d'amendement du Sénat. Quel

Cet amendement vise à permettre le bon déroulement du travail législatif. Les délais extrêmement courts entre l'examen en commission d'un projet ou d'une proposition de loi et la tenue de la séance publique, parfois cinq à six jours plus tard, rendent très difficile le travail d'amendement sur le texte de la commission. Ce qui est déjà difficile pour les membres de la commission devient encore plus compliqué pour les parlementaires qui n'en sont pas membres.

Nous proposons donc, par cet amendement, de fixer un délai raisonnable pour permettre l'exercice réel et non contraint du droit d'amendement. Quel Nous considérons que cette disposition n'est pas praticable. En effet, quand la conférence des présidents fixe le délai limite de dépôt des amendements, elle ne peut connaître la date à laquelle le texte de la commission sera adopté. Si nous adoptons ce genre d'amendement, nous risquons tout simplement de ne pas être en mesure

de deux minutes et demie. Or nous voulons laisser une chance aux collègues qui parviendraient à expliquer leur vote en moins de deux minutes et demie ! C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas suivi, malgré un élan du coeur qui l'aurait spontanément porté à le faire, la proposition de notre collègue, le président Sueur.

parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à sécuriser les parcours professionnels des collaboratrices et collaborateurs parlementaires, en valorisant l'expérience née de leur parcours professionnel. professionnel. Lors du débat sur la loi dite « de moralisation de la vie publique », dont le titre a évolué en cours de route, un amendement avait été adopté, à l'unanimité, par le Sénat,

du Sénat, en 2009 ? Le règlement du Sénat ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Y intégrer une telle exigence permettrait, enfin, de reconnaître le travail de femmes et d'hommes qui, par leur engagement professionnel

inscrite dans les instructions générales du bureau -est très défavorable aux petits groupes ou, du moins, aux groupes minoritaires. Les groupes les plus « prisés » sont rapidement choisis par les groupes majoritaires, tandis que les autres se partagent les restes. Cela n'est pas juste, un gage d'efficacité. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à modifier la règle en cours en assurant un nouveau mode de désignation des présidents des groupes d'amitié, qui laisse une plus grande place aux groupes minoritaires. Nous proposons que chaque groupe effectue le choix d'une présidence à tour de rôle, dans l'ordre de leur importance proportionnelle. Nous proposons aussi de supprimer les vice-présidents au sein des groupes régionaux, en espérant éviter ainsi, à l'avenir,

de changer les présidences, sauf au nom d'une exigence qui s'impose du fait de l'application mathématique de la règle proportionnelle. Pour des raisons

commission, modifié. En application du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, la résolution que le Sénat vient d'adopter sera soumise, avant sa mise en application, au Conseil constitutionnel. Mes chers collègues, par courrier en date de ce jour, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, a demandé que le projet de loi autorisant l'approbation des accords sur la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Suisse, d'une part, et entre la France et le Luxembourg, d'autre part, inscrit à l'ordre du jour du jeudi 20 juin, au matin, soit examiné en séance publique selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée. Acte est donné de cette demande. Dans la discussion générale, nous pourrions attribuer un temps de 45 minutes aux orateurs des groupes. Le délai limite pour les inscriptions de parole serait fixé au mercredi 19 juin à quinze heures. Y a-t-il des observations ? ? ... Il en est ainsi décidé. En conséquence, par courrier en date de ce jour, le Gouvernement demande d'inscrire à l'ordre du jour du 20 juin, au matin, l'examen de ce projet de loi en procédure normale, puis l'examen en nouvelle lecture de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires et les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de cette agence. agence. La suite de l'examen de ces textes, ainsi que du projet de loi de transformation de la fonction publique, aurait lieu après les questions d'actualité au Gouvernement. Acte est donné de cette demande. de cette demande. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique

La fonction publique est au coeur de notre pacte républicain. Elle est un maillon indispensable à la cohésion de notre société. La fonction publique, ce sont 5,5 millions d'agents publics. Près de neuf agents sur dix sont au contact direct et quotidien avec des usagers. Chaque jour, ils accueillent, accompagnent, conseillent et répondent aux attentes des Français, partout sur le territoire. Ces agents, nous les croisons tous les jours : dans les mairies, dans les écoles, dans nos hôpitaux. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, nous devons à l'ensemble de ces agents publics toute notre reconnaissance. Nous savons à quel point ils sont attachés à leurs missions et ont à coeur de rendre un service public de qualité. Puisque nos services publics tiennent une place centrale dans la société, il est de notre responsabilité d'améliorer leur accessibilité et leur efficacité. En ce sens, nous voulons donner des libertés nouvelles et accorder plus de souplesse, plus de flexibilité aux administrations pour qu'elles puissent se transformer, tant les contraintes administratives se sont accumulées. J'ai eu l'occasion d'entendre de nombreuses inquiétudes concernant nos services publics et leur réactivité. À chacun de mes déplacements dans les départements, que je parcours à raison d'une ou deux fois par semaine depuis plus de dix-sept j'ai eu l'occasion de rencontrer des employeurs publics, des élus et des encadrants, très mobilisés, soucieux de bien faire, qui m'ont souvent fait part de leur exaspération face au trop-plein de réglementations ou de cloisonnements administratifs, dont ils considèrent, à juste titre, qu'ils sont autant d'écueils qui enferment et entravent leur action. J'ai aussi rencontré des Français de toutes les générations et de tous les milieux, qui, quel que soit le territoire où ils vivent, m'ont fait part de leurs observations sur l'administration, mais aussi de leur fort attachement à leurs services publics du quotidien. Tous ces témoignages traduisent en réalité une même ambition : la recherche d'un service d'une plus grande efficacité. Réconcilier les attentes des agents, des responsables publics et des usagers, tout en renouant avec la promesse républicaine d'un service public pour tous : tel est l'objectif du Gouvernement avec ce projet de loi aujourd'hui. C'est fort C'est fort de cette volonté que nous avons voulu, avec ce texte, donner à l'ensemble des agents publics, comme à leurs employeurs, les moyens de s'adapter aux exigences contemporaines auxquelles sont aujourd'hui confrontées nos administrations. Nous souhaitons offrir aux employeurs publics de nouveaux outils de gestion des ressources humaines et d'évolution des organisations de travail. Nous voulons donner aux agents publics de nouveaux droits en matière de formation et de parcours professionnels, afin de mieux reconnaître leur engagement professionnel et de les accompagner dans leurs missions au quotidien. Ce projet de loi s'inscrit aussi dans un contexte connu de tous, celui du grand débat voulu par le Président de la République. Nous avons tous entendu, au cours de cette période, l'insatisfaction accumulée, parfois aussi la colère, de certains de nos concitoyens, lesquelles se traduisent, entre autres, par une demande de plus de proximité, couplée à une exigence de plus de solidarité. Ce besoin de plus d'égalité et de plus de justice sociale, le Premier ministre a eu l'occasion de le réaffirmer lors de son discours de politique générale prononcé mercredi dernier devant l'Assemblée nationale et ici, jeudi, lors du débat ayant suivi cette déclaration.

des Français. Ce projet de loi répond aussi, bien évidemment en partie, aux attentes qui se sont exprimées lors de cette période inédite. L'État doit donc s'adapter et être accessible à tous les citoyens, sans distinction. Pour cela, il faut des agents sur le terrain, au plus près de nos concitoyens, pour leur apporter des solutions. C'est le sens de la nouvelle étape de déconcentration que nous voulons mener. Nous avons également la volonté de repenser la localisation des services, en réinvestissant les territoires ruraux et périurbains. et périurbains. Ce texte prévoit d'apporter des solutions, des outils, pour accompagner ces mouvements et ces réorganisations. Au regard de ces exigences et d'une certaine forme d'impatience qui a pu aussi parfois se manifester, il nous faut apporter des réponses et faire en sorte que le changement soit perceptible rapidement. Il s'agit de raffermir, et même de renouveler, le lien de confiance entre nos concitoyens et nos administrations en proposant des services qui s'adaptent plus rapidement à leurs besoins et à leurs modes de vie. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi a fait l'objet d'une année entière de concertation. J'ai conduit pendant treize mois, à la demande du Premier ministre, les concertations nécessaires avec les représentants des neuf organisations syndicales de la fonction publique et avec l'ensemble des employeurs publics des trois fonctions publiques. Quatre chantiers ont ainsi été ouverts à la concertation : premièrement, le dialogue social, avec la volonté de le simplifier et de le concentrer sur l'essentiel, tout en garantissant les droits individuels et collectifs des agents l'élargissement des conditions de recrutement sous contrats, afin de permettre à nos administrations de s'adjoindre plus facilement les compétences dont elles ont besoin, et pour le temps nécessaire, tout en améliorant les conditions d'emploi des contractuels

Un cinquième chantier a pris la forme d'une négociation, qui s'est conclue le 30 novembre 2018 par la signature d'un protocole d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, avec le soutien de sept des neuf organisations syndicales représentatives et de l'ensemble des représentants des employeurs publics. Ces concertations, qui se sont achevées en février par la consultation des conseils supérieurs des trois versants de la fonction publique et du Conseil commun de la fonction publique, sont autant de moments qui nous ont permis de construire ce projet de loi équilibré. projet de loi a aussi été soumis au Conseil national d'évaluation des normes, qui a rendu un avis favorable. Je m'en félicite, car, élu local comme beaucoup d'entre vous, j'ai évidemment à coeur de respecter les collectivités et leur libre administration en matière de gestion de la fonction publique territoriale.

Il en est ainsi de la consécration du rôle du conseiller syndical, de la mise en oeuvre d'un accès renforcé à la formation pour les agents les moins bien formés ou occupant des postes présentant des risques d'usure professionnelle, ou encore, à titre d'exemple, du renforcement de certaines dispositions sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

Si l'on ne prend pas en compte les amendements visant à supprimer des articles, qui visent à rappeler des positions de principe, plus de la moitié des amendements a été retenue ou a trouvé une suite dans les travaux réglementaires que nous nous sommes engagés Pendant cette même période, j'ai reçu à de nombreuses reprises l'ensemble des associations nationales d'élus, en lien avec ma collègue Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Nous avons aussi participé à la formation, grâce à l'action de Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, de ce qui est aujourd'hui la Coordination des employeurs territoriaux. Ces derniers ont ainsi pu porter, lors de l'examen du projet de loi devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l'extension du recours au contrat pour les emplois de catégorie B. Nous assumons pleinement une forme de coconstruction avec les employeurs territoriaux, ce qui explique que certaines dispositions que nous proposons n'aient pas la même portée ou la même application dans la fonction publique territoriale et dans les deux autres versants de la fonction publique. L'enrichissement du texte s'est poursuivi lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, au cours duquel nous avons été attentifs aux propositions des députés de la majorité bien sûr, mais aussi aux positions et aux demandes exprimées par les autres groupes. Plusieurs dispositions ont ainsi été votées à l'unanimité, ou presque, des groupes parlementaires. Finalement, le texte a été adopté avec une très large majorité. Je me réjouis notamment- j'aurai l'occasion d'y revenir -que les travaux à l'Assemblée nationale aient permis de conforter le texte sur la lutte contre les situations de précarité dans la fonction publique, avec notamment la mise en place, à partir de 2021, d'une indemnité de fin de contrat pour les CDD de courte durée, à l'instar des dispositions applicables dans le secteur privé. Des changements importants ont également été apportés en matière de déontologie et d'exemplarité de la fonction publique. Je pense à la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, à l'encadrement des dispositions relatives aux nominations et aux rémunérations des présidences des autorités administratives et publiques indépendantes, ou encore à la transparence sur les plus hautes rémunérations de la fonction publique. Ce travail se poursuit désormais au Sénat. C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance des nombreux amendements adoptés en commission des lois il y a quelques jours.

Cet équilibre est fondamental si nous voulons faire adhérer agents et employeurs publics à la réforme. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que ces dispositions soient de nouveau débattues en séance, et je veillerai à vous apporter les réponses aux questions que peuvent susciter certaines d'entre elles parmi vous. Avant de détailler les mesures de ce texte, je profite de mon intervention pour réaffirmer un point essentiel, comme je l'ai déjà fait à l'Assemblée nationale : en aucune façon, ce texte ne constitue une remise en cause du statut de la fonction publique, comme j'ai parfois pu l'entendre. Le Gouvernement reste fortement attaché au statut général de la fonction publique issu de la loi de 1983, qui nous semble être un cadre essentiel pour assurer la loyauté, la compétence et l'indépendance des agents publics. En tant qu'élu local et ancien employeur public, je l'ai dit, je sais combien les enjeux sont grands et les besoins de protection des acquis des agents publics réels. Mais je sais aussi combien sont importants les besoins concrets d'adaptation du cadre de gestion de la fonction publique. C'est à cette adaptation que nous travaillons. Ainsi, nous avons veillé à ce que les dispositions fondamentales du statut général soient respectées, comme le principe selon lequel les emplois permanents de l'administration sont occupés par des agents titulaires, comme le prévoit l'article 3 de la loi de 1983, ou encore le droit à la participation des agents, par l'intermédiaire de leurs représentants, aux décisions qui les concernent. Le Conseil d'État, dans son avis, a souligné que nous avions respecté ces droits fondamentaux. Notre volonté de moderniser le statut, de le rénover, de l'adapter pour lui permettre de rester ce cadre général, protecteur et souple, de l'action de l'ensemble des agents publics est la preuve de l'attachement que nous lui portons. Par ailleurs, je souligne que ce n'est pas la première fois que le statut sera modifié ; les lois de 1983, 1984 et 1986 ont déjà connu plusieurs dizaines de modifications. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à envisager la codification des textes relatifs à la fonction publique pour en améliorer la lisibilité et l'intelligibilité. Avec ce projet de loi, nous franchissons, je pense, une nouvelle étape de la modernisation du statut et de son adaptation à la société et à ses attentes. Permettez-moi désormais de présenter plus en détail les dispositions contenues dans ce projet de loi, structuré autour de cinq titres qui sont autant de leviers de modernisation. Le premier titre simplifie les conditions d'exercice du dialogue social, pour que celui-ci soit plus stratégique, plus efficace et plus réactif, dans le respect des garanties des agents publics. projet de loi procède ainsi à une simplification de l'organisation des différentes instances de dialogue- il en existe 22 000 aujourd'hui, à l'échelle des trois versants de la fonction publique ! -, pour une plus grande déconcentration des décisions individuelles et un recentrage de ces instances sur les questions les plus qualitatives pour les agents. Ces nouvelles dispositions vont donner aux employeurs publics et aux encadrants plus de liberté en leur permettant de choisir directement les compétences dont ils ont besoin, mais aussi plus de responsabilités, nous le souhaitons, en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels pour améliorer, à leur niveau, les déroulements de carrière de leurs agents. Pour être plus précis, les décisions de mutations et de promotions ne seront plus examinées en commissions administratives paritaires, ce qui permettra de rapprocher la décision du terrain, mais aussi de gagner du temps, notamment dans l'affectation des agents publics. Pour les agents qui s'estimeraient lésés, voire discriminés, dans le traitement de leurs demandes, des voies de recours spécifiques seront mises en place. Leurs droits seront ainsi toujours garantis, et même renforcés. Nous aurons l'occasion de débattre de ce point particulier. La nouvelle instance unique, issue de la fusion du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, permettra d'aborder ensemble les questions relatives aux services, aux politiques en matière de ressources humaines et aux conditions de travail, et non plus de manière cloisonnée comme aujourd'hui. Cette instance aura à définir les règles de portée générale pour l'ensemble des sujets intéressant les relations collectives de travail, comme l'accessibilité et la qualité des services rendus, ou encore les politiques en matière de mobilité et de promotion, au regard de la gestion prévisionnelle des ressources humaines des corps et des cadres d'emploi concernés. Cet équilibre entre liberté et responsabilité est au coeur du projet de loi, et il est fondamental pour transformer la gestion des ressources humaines publiques. Dans ce même esprit, nous souhaitons développer les pratiques de négociation et permettre que des accords majoritaires puissent être conclus à l'échelon local, indépendamment de l'existence ou non d'un accord national. C'est un levier important pour responsabiliser l'ensemble des acteurs du dialogue social. Il nous semble être de nature à améliorer significativement les conditions de travail, par exemple sur des sujets comme la formation, le télétravail, l'égalité professionnelle ou encore la protection sociale complémentaire. Nous considérons que c'est en donnant plus de place au dialogue social de proximité que nous pourrons renforcer les collectifs de travail et la qualité de vie au travail. C'est la raison pour laquelle je défendrai devant vous un amendement de rétablissement de l'article 5, lequel prévoit d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur la déconcentration du dialogue social, afin de permettre des accords majoritaires locaux. Ensuite, le deuxième titre du projet de loi offre plus de souplesse aux élus et aux encadrants publics pour recruter par voie de contrat, tout en améliorant les conditions d'emploi des agents contractuels. Cette ouverture du recours au contrat a été adoptée à l'Assemblée nationale, en contrepartie de garanties renforcées en matière de transparence et de lutte contre la précarité. Pour mémoire, près de 20 % des 5,5 millions d'agents publics millions d'agents publics sont d'ores et déjà recrutés de manière contractuelle et, en flux, plus des deux tiers des recrutements se font aujourd'hui par voie de contrat, y compris dans les catégories B et C, dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas toujours satisfaisantes, ni en termes de sécurité juridique pour les employeurs ni en termes de conditions d'emplois pour les intéressés. Sans remettre en cause le principe d'occupation des emplois permanents par des agents titulaires, auquel j'ai dit notre attachement, cet élargissement du recours au contrat permettra à la fois de répondre aux besoins de compétences exprimés par les services et d'offrir des conditions d'emploi plus attractives pour les personnes qui souhaitent s'engager, pour une durée déterminée ou non, pour le service public. Sera désormais permise la nomination de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sur les emplois de direction des trois versants de la fonction publique. Cette ouverture des viviers permettra une diversification de l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique et offrira aux contractuels déjà en poste dans l'administration- je pense notamment à ceux qui bénéficient d'un CDI -de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle. Par ailleurs, un contrat de projet sera créé dans les trois versants de la fonction publique. Ce nouveau contrat permettra de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou de missions spécifiques s'inscrivant dans une durée fixée préalablement et comprise entre un an et six ans. Il sécurisera le recrutement de l'agent contractuel pour la durée du projet, tout en lui offrant des garanties en cas de non-réalisation du projet ou de fin anticipée. Au sein de l'État, le projet de loi, tel qu'il est présenté par le Gouvernement, va plus loin en généralisant à l'ensemble des établissements publics administratifs la possibilité de recourir au contrat pour l'ensemble de leurs emplois publics, à l'instar des règles qui existent aujourd'hui pour certains de ces établissements. Cette autonomie de gestion, qui nous semble nécessaire à l'exercice de leurs missions, ne fera pas obstacle à l'affectation de fonctionnaires dans ces mêmes établissements. L'article 24 du projet de loi simplifie d'ailleurs la mobilité des fonctionnaires vers ces établissements. Je sais que nous aurons à rediscuter de ce point au cours de nos débats. Cette plus grande ouverture au contrat s'accompagne aussi bien évidemment d'une professionnalisation du recrutement- tel est l'objectif de l'article 6 du projet de loi -et de garanties nouvelles en matière de lutte contre la précarité. D'une part, nous voulons lutter contre le recours abusif à la vacation dans le cadre des missions nécessitant un service à temps non complet dans la fonction publique territoriale. Je pense par exemple au temps d'accueil périscolaire ou aux personnels de cantine. Plusieurs options seront désormais offertes aux employeurs publics pour répondre à ces besoins : recrutement par voie de contrat, recrutement titulaire, recours au centre de gestion, qui exercera alors un rôle de « groupement d'employeurs », de manière à lutter contre la précarité et à sécuriser agents et employeurs. D'autre part, la prime de précarité, introduite à l'Assemblée nationale à la demande de la majorité, permettra aux agents publics de bénéficier des mêmes garanties que les salariés de droit privé, tout en tenant compte de la gestion spécifique des contrats dans la fonction publique. sera-t-elle réservée aux contrats d'une durée inférieure ou égale à un an, soit 70 % des contrats conclus, prévoyant une rémunération n'excédant pas deux SMIC, soit 3 000 euros bruts par mois. Ce dispositif entrera en vigueur pour les contrats conclus à partir de 2021, de manière à laisser le temps aux employeurs publics de s'approprier les nouveaux leviers prévus dans le projet de loi. Pour information, à pratiques de recrutement inchangées, le coût du dispositif s'élèverait à environ 350 millions d'euros par an, tous versants confondus, dont environ 150 millions d'euros pour la fonction publique territoriale. Il est essentiel que ce dispositif bénéficie dans les mêmes conditions aux agents des trois versants de la fonction publique. Je défendrai donc devant vous deux dispositifs conjuguant le rétablissement de l'intégralité de cette mesure, tout en tenant compte de la situation spécifique de la fonction publique hospitalière, qui présente des besoins particuliers.

par une plus grande responsabilisation des employeurs publics, qui peuvent s'appuyer, depuis 2016, sur un référent déontologue. Un nouveau contrôle est également mis en place, à l'entrée dans la fonction publique ou au retour de mobilité dans le secteur privé, pour les personnes nommées à des emplois de direction.

totalement indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions. Ce nouvel équilibre nous paraît essentiel pour préserver la prise en compte des spécificités du cadre de gestion des agents publics, sachant que la nouvelle HATVP aura à connaître des règles de portée générale, mais aussi d'un grand nombre de situations individuelles dans chacun des versants de la fonction publique et des dispositifs spécifiques dont bénéficient les chercheurs au titre du code de la recherche. En termes d'exemplarité, de nouvelles règles ont été introduites à l'Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, s'agissant des rémunérations de la haute fonction publique transparence des dix plus hautes rémunérations au sein de chaque administration, collectivité et établissement de santé, et rapport annuel au Parlement. Par ailleurs, les rémunérations des présidents et membres des autorités administratives et publiques indépendantes seront encadrées et plafonnées en cas de cumul avec une pension de retraite. En matière d'équité, le projet de loi met fin aux dérogations existantes en matière de durée légale du travail, soit 1 607 heures, sauf sujétions particulières comme le travail de nuit, le week-end ou les jours fériés, ou les travaux pénibles. Les accords dérogatoires à la loi de 2001 en vigueur dans la fonction publique territoriale devront être supprimés au plus tard un an après le renouvellement des assemblées délibérantes. Nous aurons l'occasion de rediscuter de ce délai. Au sein de l'État,

C'est aussi au titre de la transparence et de l'équité entre les agents publics que ce projet de loi prévoit, dans le prolongement du rapport de MM. Jacques Savatier, député, et Arnaud de Belenet, sénateur- je les salue et les remercie de nouveau pour leur travail de nouveaux leviers pour améliorer la qualité du service rendu par le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. L'objectif est d'améliorer la coopération et les mutualisations entre les centres de gestion, d'une part, et entre les centres de gestion et le CNFPT, d'autre part, à l'échelle de chaque région. Il s'agit aussi de renforcer la transparence sur l'utilisation des crédits dont bénéficie le CNFPT et de lui permettre de mettre en oeuvre les obligations prévues par le législateur, notamment le financement du développement de l'apprentissage, au bénéfice de toutes les collectivités territoriales.

C'est aussi dans cette partie du projet de loi que nous prévoyons la possibilité, par voie d'ordonnances, d'améliorer les conditions de travail des agents publics, de renforcer et d'harmoniser leurs droits en matière de protection sociale et de mieux prévenir et mieux traiter les situations d'inaptitude physique dans la fonction publique. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que rencontrent aujourd'hui un grand nombre d'employeurs publics pour garantir la santé et la sécurité au travail de leurs équipes. Des travaux ont déjà été engagés sur les questions de protection sociale complémentaire, d'accès à la médecine de prévention et d'accompagnement individuel des situations de reclassement. Il nous faut aller plus loin. C'est l'ambition du Gouvernement. Nous attendons les conclusions de la mission parlementaire en cours, conduite par la députée Charlotte Lecocq, pour lancer les travaux de concertation complémentaires. De la même manière, nous nous appuierons sur les conclusions de la mission de M. Frédéric Thiriez sur le recrutement et la gestion des carrières dans la haute fonction publique, prévues pour novembre prochain, avant d'engager la concertation sur les évolutions à apporter, ces enjeux étant aussi très importants pour l'avenir et l'attractivité J'en viens maintenant au quatrième axe du projet de loi. Il s'agit de décloisonner les carrières en permettant une plus grande mobilité entre les versants de la fonction publique, mais aussi entre les secteurs public et privé, tout en accordant plus de sécurité, de droits et d'accompagnement pour les agents concernés. Tout d'abord, nous souhaitons l'introduction d'un mécanisme de rupture conventionnelle, afin de favoriser la réalisation de projets d'évolution professionnelle des agents publics en leur donnant les mêmes garanties qu'aux salariés : le bénéfice d'une indemnité de rupture et de l'assurance chômage. Ces dispositions seront applicables aux agents en CDI et, à titre expérimental, aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique. Par ailleurs, le projet de loi renforce les garanties applicables aux agents publics en cas de restructuration. notamment, et c'est une nouveauté, la garantie d'être affectés à un nouvel emploi dans le département dans lequel ils exercent leurs fonctions, le bénéfice d'un congé de transition professionnelle rémunéré pour changer de métier et se former à un nouveau poste, une indemnité de départ renforcée, avec le bénéfice de l'assurance chômage, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre

j'en viens au cinquième axe, le renforcement de l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Le projet de loi met en oeuvre les engagements que nous avons pris collectivement dans le cadre de l'accord majoritaire du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s'agit d'instaurer des plans d'action pour traiter notamment des problématiques d'écarts de rémunération, de renforcer le dispositif de nominations équilibrées aux emplois de direction, de ne plus appliquer le jour de carence pour maladie aux agents en situation de grossesse, ou encore, comme pour les agents de l'État, de garantir le maintien des primes et des indemnités versées par les collectivités territoriales pour les agents durant les congés pour maternité,

et l'élargissement du champ des handicaps pris en compte, la suppression de la référence au handicap physique, pour pouvoir bénéficier d'aménagements d'épreuves lors des concours, par exemple. Ces dispositions s'ajoutent à la rénovation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mise en oeuvre par la loi son avenir professionnel, portée par ma collègue Muriel Pénicaud, qui va permettre de simplifier le recrutement de personnes en situation de handicap, notamment dans les structures à faibles effectifs, et de renforcer la capacité d'action du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, en sécurisant son financement d'ici à trois ans. J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du récent rapport du Sénat sur la politique du handicap dans la fonction publique, rédigé par Catherine Di Folco et Didier Marie. Le Gouvernement est ouvert aux amendements visant à enrichir le texte et à renforcer les garanties offertes aux agents publics en situation de handicap, dans le respect

Madame la présidente, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, d'autres chantiers de modernisation de la fonction publique sont en cours et les concertations se poursuivent. Je pense notamment à la question de l'attractivité des concours de la fonction publique ou encore à la préparation du rendez-vous salarial programmé le 2 juillet prochain.

J'en suis convaincu, les débats des prochains jours ne manqueront pas d'enrichir notre réflexion collective, ainsi que le projet de loi lui-même. Ce projet de loi simplifie la gestion des ressources humaines, en tenant compte des spécificités de chaque versant et comprend des avancées fortes pour améliorer le quotidien des agents publics. C'est dans l'intérêt de nos concitoyens que nous vous soumettons ce projet de loi de transformation de la fonction publique. Il s'agit de renouer avec la promesse républicaine d'un service public pour tous, en apportant, par des mesures concrètes et opérationnelles, une plus grande qualité de service, notamment dans les territoires les plus reculés, mais aussi d'offrir aux agents et aux cadres de la fonction publique, qui s'engagent au quotidien, un meilleur environnement de travail et des perspectives nouvelles d'évolution professionnelle. Vous l'avez constaté, le Gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements.

Son intitulé paraît quelque peu ambitieux, car il s'agit non d'une véritable transformation de la fonction publique, mais plutôt d'une série de modifications, souvent techniques, pour une fonction publique « plus agile En préambule, Loïc Hervé, également rapporteur de ce texte, et moi-même saluons le travail de ces femmes et de ces hommes qui oeuvrent au quotidien pour la bonne organisation des services publics. La fonction publique constitue, en effet, notre bien commun, qu'il convient de préserver, tout en modernisant son organisation pour l'adapter aux nouveaux besoins des employeurs publics et aux nouveaux métiers.

Les représentants des employeurs publics ont, en revanche, soutenu les principaux objectifs du projet de loi, montrant un intérêt particulier pour les nouveaux leviers de gestion des ressources humaines. Nous avons également lancé une consultation en ligne à l'attention des employeurs territoriaux, laquelle a remporté un vif succès. Ainsi, 2 200 élus locaux ont donné leur avis, 42 % d'entre eux représentant des communes de moins de 1 000 habitants. Les principales attentes des employeurs territoriaux concernent la reconnaissance des performances professionnelles des agents, la simplification du dialogue social et l'élargissement du recours aux agents contractuels. Bien qu'il ne traduise pas une réelle vision de l'action publique, ce projet de loi comporte une palette d'outils permettant une meilleure gestion des ressources humaines. Nous avons donc adopté une attitude pragmatique tendant à élargir cette palette tout en respectant les droits des agents publics et les grands principes du statut général. La commission des lois a adopté 154 amendements visant trois objectifs : tout d'abord, préserver les spécificités de la fonction publique territoriale et mieux répondre aux attentes des employeurs locaux mieux reconnaître le mérite des agents et garantir leurs droits ; enfin, encadrer plus précisément la réforme de la haute fonction publique, afin de garantir son excellence tout en renforçant sa diversité. Afin de mieux répondre aux attentes des employeurs territoriaux, la commission des lois a souhaité donner plus de prévisibilité aux élus locaux. L'État aurait désormais l'obligation de publier une feuille de route triennale dans laquelle il indiquerait l'incidence financière de ses décisions en matière de ressources humaines sur les budgets locaux- c'est ce que prévoit La commission a supprimé un renvoi à un décret en Conseil d'État pour préciser les fonctions exercées par le directeur général des services, renvoi qui constituerait une atteinte grave à la libre administration des collectivités territoriales. De même, à l'article 7, la liberté de recrutement des employeurs territoriaux a été réaffirmée, dans le respect du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics. La commission des lois a souhaité accorder davantage de souplesse, notamment, à l'article 10, en permettant aux communes de moins de 2 000 habitants de pourvoir l'ensemble

les employeurs territoriaux disposeraient de dix-huit mois à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour organiser la concertation sur l'harmonisation du temps de travail, contre douze mois dans le projet de loi initial.

adoptée par l'Assemblée nationale, le projet de loi permettait un recours aux agents contractuels plus étendu dans la fonction publique d'État que dans les deux autres versants. La commission des lois a souhaité rétablir un certain équilibre à l'article 9 en supprimant, dans le versant étatique, l'extension du recours au contrat pour les emplois des établissements publics à caractère administratif, ainsi que pour les emplois

la commission s'est préoccupée des 3 000 fonctionnaires appartenant aux corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française, les CEAPF. Pour faciliter la promotion interne de ces agents, le nouvel article 33 prévoit la création des corps de catégorie A au sein des CEAPF.

À défaut de faire révolution, ce texte comprend de nombreuses dispositions qui vont dans le bon sens et qui consacrent souvent des évolutions déjà en cours dans nos fonctions publiques. En complément de l'intervention de ma collègue rapporteur, j'aborderai divers domaines, notamment la réforme de la haute fonction publique. La commission des lois a souhaité préciser, par conséquent restreindre, le périmètre de l'habilitation à légiférer par ordonnance. Quelle idée ! En effet, sur ce point, de se fonder sur les travaux de la mission confiée par le Président de la République et le Premier ministre à maître Frédéric Thiriez en privilégiant un tronc commun d'enseignements des écoles de services publics. À ce stade, la fusion de plusieurs de ces écoles ne me semble ni souhaitée ni souhaitable. Venons-en à la déontologie : si la plupart des freins à la mobilité des fonctionnaires sont levés,

Concernant les avis, la commission des lois a fait le choix, plus respectueux des libertés publiques, de laisser à la discrétion de la HATVP la décision de leur publication. Nous avons également souhaité contraindre explicitement la HATVP à prendre en considération la carrière des agents concernés, afin de favoriser une véritable politique de ressources humaines dans les plus hautes sphères de l'État. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a aussi été renforcée par plusieurs mesures. D'une part, un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissement sexiste a été instauré. D'autre part, le texte de la commission étend l'obligation de nominations équilibrées dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique en élargissant le champ des emplois et des administrations concernées. D'autres correctifs ont été apportés, comme l'exemption du jour de carence pour les femmes enceintes et le maintien des droits à avancement des agents bénéficiant d'un congé parental. Les droits sanitaires et sociaux des agents ont été renforcés. Au-delà de l'amélioration de l'intégration des agents en situation de handicap, sujet abordé par Catherine Di Folco, le congé du proche aidant sera étendu à l'ensemble de la fonction publique, ce qui permettra aux agents d'apporter leur aide à un proche souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Par ailleurs, les femmes fonctionnaires pourront bénéficier d'une heure par jour pour allaiter leur enfant, disposition déjà en vigueur dans le secteur privé. Enfin, il était primordial de doter la fonction publique territoriale de moyens pour développer l'apprentissage, depuis la perte de compétence des régions en matière d'aides financières aux employeurs territoriaux. Nous souhaitons donc que l'État participe à hauteur de 23 millions d'euros au financement de l'apprentissage. Monsieur le secrétaire d'État, vous l'aurez compris, le Sénat a fait oeuvre utile en enrichissant le projet fidèle à la mission que lui assigne la Constitution, en améliorant la loi, en intégrant dans le texte ses travaux les plus récents, en représentant les territoires et les besoins de nos concitoyens, afin de leur donner une fonction publique à la hauteur des enjeux de notre temps.

texte très important, qui touche au coeur du pacte républicain, puisqu'il s'agit des conditions de travail de celles et de ceux qui font vivre au quotidien les services publics. Infirmières, médecins, gendarmes, juges, enseignants, chercheurs, bibliothécaires, agents territoriaux, personnels de crèche et des écoles, cantonniers je veux, au nom de mon groupe, leur rendre hommage. Quotidiennement, dans des conditions difficiles faites de coupes budgétaires, de perte du pouvoir d'achat et de défiance parfois, ces

Ce gouvernement, comme les précédents, n'a qu'une boussole, pour ne pas dire qu'une obsession : baisser la dépense publique, réduire l'action de l'État, laissant ainsi la place aux marchés financiers et aux intérêts privés. Il s'agit au fond de lever tous les obstacles pour déréguler et libéraliser. Pour ce faire, tout est bon des budgets dans les lois de finances successives, baisse des dotations pour les collectivités, externalisation et privatisation à tout crin. Aujourd'hui, avec ce projet de loi, l'État se lance dans une nouvelle étape sur le chemin de la privatisation.

en cohérence d'ailleurs avec les objectifs fixés par le rapport CAP 2022 et les ordonnances récentes du Premier ministre sur la réorganisation de l'État. Le cap est cohérent, puisqu'il s'agit encore et toujours d'accentuer les transferts de charges et d'abandonner des services faute de rentabilité suffisante. On gère l'État comme une entreprise. Si seulement ! C'est l'avènement de la start-up nation. Pour justifier ces politiques de reculs sociaux, le Gouvernement joue la carte dangereuse du tous contre tous, faisant passer les fonctionnaires pour des privilégiés, et ce alors même que la majorité d'entre eux, comme les gilets jaunes, ont du mal à boucler leurs fins de mois au regard des salaires extrêmement bas dans la fonction publique. Voilà la réalité, mes chers collègues Ce texte organise ainsi une remise en cause totale des règles fondamentales de l'organisation des pouvoirs publics, donc de la fonction publique. Il remet en question le statut établi à la sortie de la guerre, en 1946, pour créer une fonction publique aux ordres non pas d'une hiérarchie potentiellement arbitraire et autoritaire, voire antirépublicaine, mais bien de l'intérêt général. Doit-on rappeler cela aujourd'hui, en ce jour anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle ?

plaçant le fonctionnaire dans une distance juste par rapport à sa hiérarchie, lui permettant même de désobéir à des ordres illégaux. Les lois Le Pors de 1983 et 1984 ont conforté ce statut accompagnant notamment la décentralisation, des innovations majeures qui ont permis d'établir un statut à la fois souple et solide. Trois principes ont présidé à cette construction et au socle de ce statut. Premier principe, le

formule ! Ainsi, seul le concours permet, en droit, d'assurer l'égalité d'accès des citoyens à la fonction publique. Deuxième principe, le principe d'indépendance, qui conduit à distinguer le grade, propriété du fonctionnaire, de l'emploi, à la disposition de l'administration.

qui dispose : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Il s'ensuit que le fonctionnaire, parce qu'il est soumis à cette obligation de service du bien commun, doit avoir la plénitude des droits et devoirs du citoyen et non être regardé comme le sujet du pouvoir politique ou le rouage impersonnel de la machine administrative. Ces trois principes, ainsi que la stabilité de l'emploi public, le mal nommé « emploi à vie », permettent de garantir que les agents des services publics soient indépendants et libres par rapport aux forces politiques et aux forces de l'argent. Ce sont ces règles qui protègent du clientélisme et de la corruption, qui gangrènent tant de systèmes politiques. En appliquant le modèle des ordonnances de la loi Travail à la fonction publique, ce projet de loi rompt avec ces principes fondateurs, tout en attaquant en attaquant les principes de démocratie sociale. Il s'en prend tout d'abord au principe d'égalité par le contournement du concours et le recours massif aux contractuels sur des emplois permanents et de direction. Or ce dispositif, contrairement aux attendus de l'exposé des motifs, va encourager le pantouflage, voire le rétropantouflage, participant à brouiller les finalités de l'action publique. Il participe par ailleurs à une précarisation accrue des agents publics, notamment au travers du nouveau contrat de projet. Pourtant, mes chers collègues, comment ignorer que, si les agents sont précaires, le service public lui-même sera précarisé ?

Le principe d'indépendance est également remis en cause, puisque le recours au contrat favorisera l'embauche, comme aux États-Unis, d'une fonction publique aux ordres du pouvoir politique, car très directement liée à elle. Le renforcement du pouvoir hiérarchique par la remise en question des instances paritaires, mais également par la montée en puissance de la rémunération au mérite, accentuera ce phénomène, notamment au sein de la fonction publique territoriale. Avec l'ensemble de ces procédés, il s'agit au fond de placer l'agent dans un rapport individuel à l'égard de l'administration, ce qui le déconnectera de l'intérêt général et le rendra ainsi plus vulnérable aux pressions administratives, politiques ou économiques. On crée pour demain une main-d'oeuvre publique corvéable, manipulable, mutable et révocable à merci. Les maires ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en appelant dans une tribune au retrait de ce projet de loi, au nom de la cohésion sociale et territoriale de la Nation. a également fait part de ses réserves. Le mouvement des gilets jaunes a plébiscité, lui aussi, les services publics, comme leviers puissants de redistribution sociale. Vous faites tout le contraire avec ce projet de loi, en faisant prévaloir la liberté contractuelle sur l'égalité républicaine ! Par ailleurs, le Gouvernement utilise l'argument de la mobilité, non pas comme un droit, mais comme une opportunité pour encourager les fonctionnaires à quitter la fonction publique en favorisant les ruptures conventionnelles. Il accompagne la privatisation des services publics et le désengagement de l'État en prévoyant le détachement d'office des fonctionnaires. Ce projet de loi crée ainsi les outils destructeurs d'un dégraissage massif et d'une rupture de l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire. Notons pour être justes

ces miettes ne peuvent nous faire oublier l'essentiel de ce texte : le dépérissement du statut et la soumission de l'État et des pouvoirs publics aux règles de management issues du privé, donc incompatibles avec les missions spécifiques du service public. À nos yeux, les enjeux de modernisation se situaient fondamentalement ailleurs. à l'enjeu de démocratisation, afin de mieux prendre en compte les besoins au plus près des territoires et des usagers. Nous pensons aussi à l'enjeu de transition écologique- les fonctionnaires sont une richesse incroyable dans ce défi par leur adaptabilité et leur sens du temps long. Nous pensons encore à l'enjeu de rénovation des concours et des formations pour les ouvrir à la société telle qu'elle est dans sa diversité, donc dans sa richesse. Nous devons par ailleurs collectivement nous atteler à un vaste plan de reconquête sur le secteur privé, qui n'a pas la capacité, nous le constatons tous les jours, de répondre aux besoins de nos concitoyens. Pour faire face à l'ensemble de ces enjeux, notre pays n'a pas besoin de moins de fonctionnaires, ni même de fonctionnaires précarisés, pas plus que des règles de management issues du privé. Nous voyons à cet égard les conséquences dramatiques de ces méthodes à France Télécom. notre pays doit pouvoir s'appuyer sur un statut protecteur comme le corollaire de la qualité du service rendu, sur des agents enfin reconnus et valorisés. À l'heure où les dangers du repli sur soi et du rejet de l'autre n'ont jamais été aussi forts, il est urgent de promouvoir un projet permettant de créer du lien, de favoriser les communs, la solidarité et la cohésion sociale et territoriale, c'est-à-dire, au fond, de redéfinir dans le cadre du pacte républicain. Les services publics en sont le levier principal. Vous l'avez dit, la fonction publique est une richesse, le bien commun de la Nation. Oui, c'est vrai ! Il s'agit le plus souvent du premier contact de nos concitoyens avec l'État. Nous demandons, à l'instar de l'ensemble des organisations syndicales, le retrait de ce texte, qui organise une nouvelle fois l'incurie de l'État à répondre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens.

a tenu à maintenir le rôle des CAP en matière d'avancement et de promotion interne. Elle a établi un meilleur contrôle du rétropantouflage lorsqu'un agent contractuel est recruté dans un emploi de direction. a prévu l'élaboration d'une feuille de route pour mieux anticiper les décisions du Gouvernement, notamment en matière d'évolution du point d'indice. Elle a reconnu de nouveaux droits, comme le congé de proche aidant ou le droit à la portabilité pour les agents handicapés.

Il est attendu par les employeurs, qu'ils soient élus ou encadrants, qui expriment non seulement leur besoin d'autonomie et de souplesse, mais aussi leur demande de confiance. La déconcentration des décisions est le signe de cette confiance que nous voulons leur témoigner. Ce texte est également attendu par les agents. J'ai rencontré plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'agents qui m'ont fait part de leur sentiment parfois d'être assignés à résidence professionnelle, de leur volonté de trouver des perspectives dans la fonction publique ou- plus rarement, c'est vrai, mais cela arrive assez régulièrement -dans le secteur privé, et qui souhaitent avoir des outils et des sécurisations pour cela.

met gravement en cause notre pacte républicain par une attaque frontale contre les fondements de la fonction publique, donc contre les services publics. Plus précisément, à l'échelon des collectivités territoriales, les élus locaux n'étaient pas demandeurs de cette réforme. Aujourd'hui, ils la rejettent massivement. un appel des maires de toute sensibilité politique demande le retrait de ce projet de loi au nom de la cohésion sociale et territoriale : « Les maires ont besoin de fonctionnaires aux rôles et fonctions définis par un statut durable à l'image de la continuité républicaine, aux compétences validées par des diplômes et ayant réussi des concours officiels dans le cadre de référentiels nationaux, neutres politiquement, totalement voués à l'accomplissement de leurs missions de service public, quelles que soient les alternances. « Cette qualité, cette stabilité, cette indépendance des fonctionnaires sont des conditions essentielles afin de garantir pour tous et partout des services publics de haut niveau.

La création de la fonction publique territoriale, en parallèle des lois de décentralisation au début des années quatre-vingt, a été une innovation majeure au bénéfice des territoires permettant dans le même temps de garantir un haut niveau de compétence et de sécuriser les élus employeurs. Le retour de l'arbitraire est donc un très mauvais présage, y compris pour les usagers des services publics locaux, d'autant que le passage du texte en commission a renforcé non seulement la capacité de recours aux contractuels pour les collectivités, notamment dans les communes de moins de 2 000 habitants, mais également la rémunération au mérite favorisant l'inégalité entre les agents. Mes chers collègues, les collectivités ont souvent été une source d'innovation, je dirais même de créativité pour la conquête de droits nouveaux pour nos concitoyens, que ce soit pour la petite enfance, le service de l'eau, etc. Elles ont permis d'ouvrir par leurs politiques des pans de l'intérêt général. Voilà la véritable finalité d'un droit à la différenciation. Aujourd'hui, la conjugaison de la diminution des dotations et de l'injonction d'une baisse de l'emploi public porte gravement atteinte à cette capacité d'initiative, et il ne suffira pas de vouloir constitutionnaliser demain ce droit à la différenciation

en déposant des amendements de suppression d'articles. Nous sommes en effet opposés aux deux principes qui guident ce projet de loi : l'affaiblissement du dialogue social et la mise en concurrence des fonctionnaires avec les contractuels. Nous avons aussi décidé de faire des propositions, parce que nous sommes attachés à la conception française de la fonction publique. Cependant, nous partageons les préoccupations exprimées par nos collègues du groupe CRCE quant aux conséquences prévisibles de ce texte pour la fonction publique dans son ensemble. En affaiblissant comme jamais le dialogue social, à tous les étages, le Gouvernement cherche manifestement à réduire le poids des partenaires sociaux pour préparer le terrain à une restructuration et à une réorganisation majeure des trois fonctions publiques. Plusieurs milliers d'instances de dialogue vont disparaître. Cette décision porte en germe une détérioration des conditions de travail préjudiciable aux agents, mais tout autant aux employeurs. Les moyens des organisations représentant les personnels s'en trouveront fortement diminués, ce qui facilitera le passage du rouleau compresseur ayant pour mission d'aplatir la fonction publique et de la purger de 120 000 postes. En ouvrant très largement le recours au contrat, le Gouvernement n'abolit pas le statut ; il le contourne, en aggravant la précarité. Vous faites, monsieur le secrétaire d'État, le choix de la banalisation de la fonction publique et de l'affaiblissement de l'action publique. Le contrat, c'est l'antithèse d'une fonction publique de carrière. Vous prenez le risque, en faisant reculer les règles déontologiques, de la confusion entre intérêt public et intérêts privés, à la faveur du pantouflage et du rétropantouflage, au moment même où la demande de transparence n'a jamais été aussi forte.

nous étions prêts à engager le débat sur ce texte. Nous n'en avons pourtant pas eu l'opportunité, tant les conditions d'examen de celui-ci sont déplorables et relèvent d'un déni de démocratie.

Nous avons ainsi déposé des amendements, que nous défendrons avec ardeur. Nous choisirons le meilleur pour nos trois fonctions publiques, qu'il faudra parfois différencier. C'est pourquoi nous espérons que chacun s'écoutera pour construire ce texte.